La séance est reprise, nous reprenons la discussion de la mission enseignement scolaire du projet de loi de finances pour 2000 au regard du nombre d'amendements examinés en accord avec la commission des finances, nous pourrions porter à titre exceptionnel. La durée maximale prévisionnel de cette mission de 3 à 4 heures, ce qui devrait nous conduire achevé nos travaux aux alentours de 0

nous reprenons la discussion générale et la parole est à Madame Marie-Pierre Monier pour le groupe socialiste, écologiste républicains pour 9 minutes. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, dans son discours du 6 juin 1889 sur l'école laïque, Jules Ferry, déclaré que l'Havre scolaire de la IIIe République appartenait au pays républicain tout entier cet héritage d'une école publique, laïque et républicaine, nous en sommes toutes et tous, responsables, il me semble aujourd'hui qu'il est à la croisée des chemins, la crise des vocations qui. Frappe le monde enseignant cristallisés par la pénurie de candidats au concours et la recrudescence des démissions résonne comme un signal d'alarme dont il nous faut tirer les bonnes leçons les professeurs de ce pays en soif de reconnaissance de la part de l'institution et de la société en général est un des leviers de cette reconnaissance, c'est leur niveau de rémunération, rappelons que les enseignants français ont perdu entre 15 et 25 % de pouvoir d'achat en 20 ans que leur paye en début de carrière et 7 % en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, un chiffre qui monte jusqu'à 15 % après 15 ans de métier prenant acte de ce constat, le gouvernement a choisi dans la continuité de la politique menée lors du précédent quinquennat de concentrer ses efforts sur les débuts de carrière jugés prioritaires si l'effort budgétaire consenti dans ce cadre est significatif, à l'instar de la hausse des crédits pour l'ensemble de la mission enseignement scolaire programmée dans le cadre de ce PLF, il convient d'y apporter un regard critique pour plusieurs raisons l'augmentation de plus 5 82 % est inférieure à l'inflation, ensuite, elle doit être considéré, au regard de l'importance des effectifs enseignants dans leur ensemble 856500 par ailleurs le ciblage de cette revalorisation sur le début de carrière, signifie que les 42 % d'enseignants dépassant les 20 ans d'exercice seront confrontés à une nouvelle stagnation dans leur rémunération pour y remédier, il aurait proposé une accélération des promotions en fin de carrière et la souscription au fameux Pacte enseignants qui conditionne une augmentation de salaire au fait d'assumer de nouvelles missions dans la volant pas louer s'élève à 300 millions sur 935 millions consacrés à la revalorisation, c'est l'ancienne professeur de maths. Thématique qui vous parle, le raisonnement niché dans ce pacte qui sous-entend que les professeurs disposeraient aujourd'hui d'un surplus de temps libre à mettre à profit et au mieux une illusion, au pire un mensonge les chiffres des services statistiques du ministère de l'Éducation nationale sont clairs à cet égard la moitié des enseignants ont un temps de travail supérieure à 43 heures par semaine, c'est une médiane durant les 16 semaines de vacances scolaires dont ils disposent, la moitié des professeurs déclare travailler au moins de 34 jours la logique du travailler plus pour gagner plus que traduit ce pacte se heurte donc à la réalité du terrain et on ne peut que constater le flou qui persiste sur la nature de ses nouvelles missions, à l'heure où la moitié d'entre eux signalent un sentiment d'épuisement professionnel élevé comme le montre le premier bar baromètre du bien-être au travail des personnels de l'éducation nationale, la volonté du ministère, de s'engager dans cette voie apparaît d'autant plus discutable, il y a donc de nombreuses limites au choc d'attractivité mise en avant par le gouvernement, et au vu de l'évolution des crédits programmés pour la mission enseignement scolaire pour les prochaines années, les marges de manoeuvre ou pour l'accentuer apparaissent bien restreinte, par ailleurs, les attentes des enseignants porte également sur les conditions d'exercice de leur mission et à cet égard, plusieurs aspects de ce budget ne sont pas à la hauteur, je pense notamment aux suppressions de postes qui s'élève à respectivement 1117 postes dans le 1er degré et 480 dans le second degré, les suppressions de postes pour le 1er degré apparaissent en décalage avec la poursuite des politiques de dédoublement en plus en CP, CE1 et grande section et le plafonnement 24 élèves par classe dans ces mêmes niveaux hors éducation prioritaire dont nous continuons à saluer le principe d'un autre rapport sur le bilan des mesures éducatives du précédent quinquennat menée avec mes collègues ah Ligue bilan et Max Brisson, nous nous étions déjà interrogé sur l'écart entre les moyens nécessaires pour les mettre en place et les ETP effectivement créé, il manquerait 12200 pour l'enseignement secondaire, ces nouvelles suppressions s'inscrivent dans un contexte très dégradé après la suppression de 7500 postes de 2018 à 2021 alors que les effectifs ont enregistré une hausse de plus de 68000 élèves sur cette même période, dans mon département de la Drôme, les conséquences très concrète de ces suppressions se sont fait sentir, certains établissements ont fait leur rentrée après une ou plusieurs fermetures de classes, ce qui signifie des effectifs élevés et dans de moins bonnes conditions de travail pour les pour les élèves comme pour les enseignants, d'autres ont perdu des postes d'enseignement, parfois, cela signifie la fin de l'association sportive ou la disparition de l'éducation au développement durable, car les références ne sont plus là où doivent assumer d'autres missions, en ce qui concerne l'école inclusive, nous aurons l'occasion de reparler très prochainement des conditions d'emploi et de travail des accompagnants des élèves en situation de handicap à l'occasion de l'examen de la proposition de loi les concernant la semaine prochaine, l'état des lieux, qui est ressorti des nombreuses ambitions que j'ai pu mener dans ce cadre, et tout particulièrement préoccupant, modalités de recrutement dans les conditions de travail, niveau de rémunération, de formation, sont autant de chantiers à investir et je suivrai avec attention les travaux prévus dans le par le ministère à ce sujet, je salue la création de 4000 nouveaux postes d'AESH mais qui ne suffira ont néanmoins pas à répondre aux besoins créés par les notifications, ainsi que l'augmentation de 10 % de crédits alloués à la rémunération des AESH dont il convient de préciser les modalités de répartition je conclurai en évoquant l'enseignement agricole, vecteur de richesses et d'innovation pour nos territoires dans nous reconnaissant toutes et tous la valeur sur ces ben je salue la présence du ministre de l'agriculture à l'occasion de cet examen, qui témoigne de son intérêt sur le sujet, nous avons su lors de précédents exercices budgétaires nous rassembler largement pour appuyer une hausse de crédit qui lui sont consacrés, les besoins étant d'autant plus criant au regard des impératifs de transition agroécologique et de renouvellement des générations, nous ne pouvons pas nous réjouir en l'état du budget qui nous est présenté aujourd'hui, car s'il ne prévoit pas de nouvelles suppressions de postes d'enseignants, qui est une bonne chose, il ne prévoit pas non plus de créations, c'est pour moi un manque de volontarisme et cela interroge après la forte dégradation opéré sous le précédent quinquennat ou pour rappel : plus de 300 emplois ont été supprimés, ce qui, en proportion, correspondrait à une suppression de 10000 postes dans l'Éducation nationale, ces suppressions ont eu des impacts très concrets sur les conditions d'enseignement à l'instar de la fin du dédoublement obligatoire qui s'était fait opéré au détriment de la qualité de l'apprentissage et de la sécurité des élèves, si le président de la République est sincère dans sa volonté de mettre en oeuvre un parc d'orientation et d'avenir agricole alors les moyens alloués doivent être à la hauteur de cette ambition, vous l'avez compris nous, estimant que la méthode choisie pour répondre aux besoins de revalorisation salariale et à la perte d'attractivité du métier d'enseignant n'est pas adapté aux réalités, pas plus que ne l'est l'équilibre entre créations et suppressions de postes, ce budget s'inscrit dans une continuité de choix politiques qui, depuis plusieurs années ont fragilisé notre école républicaine, ce sont ces mêmes choix qui conduisent aujourd'hui à pallier des manques en utilisant une méthode libéral d'appels à projets sur le modèle de l'école du futur qui permettra seulement à certaines écoles de sortir la tête de l'eau, tandis que d'autres seront laissés sur le bord du chemin, nous craignons que notre école de la République ne soit pas renforcé par ce budget 2023 et nous voterons donc contre. Merci, cher collègue, dans la suite de la discussion, la parole est à madame Céline Brulin pour le groupe CRCE pour cinq minutes. Monsieur le président, messieurs les ministres, et je salue, à mon tour la présence du ministre de l'Agriculture parmi nous, vous présentez ce budget comme celui d'une ambition inédite en matière d'éducation mais nous en sommes malheureusement loin il manque encore un enseignant dans un tiers des établissements scolaires mais vous prévoyez la suppression de plus de 1500 postes, vous arguez la baisse démographique et promettait un meilleur taux d'encadrement, mais il existe de nombreux départements, dont le mien, où l'on compte des classes bien plus de 24 élèves or REP, alors que ce ne devait plus être le cas, à l'issue du précédent quinquennat vous annoncer la mise en place de l'école du futur ou les moyens ne serait plus allouées en fonction des besoins des élèves en fonction de critères objectifs, mais pour des projets dits innovants sans que vous n'en faisant définissiez ce concept, si ce n'est que d'améliorer la réussite des élèves, comme si, auparavant, les établissements scolaires ne travaillait pas déjà en ce sens, je crains que la communauté éducative ne se satisfasse pas de ce qui s'apparente en réalité à un exercice de communication, le cas de l'enseignement technique agricole illustre parfaitement cela une loi d'orientation agricole est prévue pour 2023, dans laquelle il est annoncé que la part de l'enseignement et de la formation se majeur, hé bien aucun projet stratégique n'est défini à ce stade, tout juste est-il mis fin à la saignée opérée ces dernières années dans l'enseignement agricole public de même, les récentes déclarations présidentielles ont confirmé la volonté politique de démanteler l'enseignement professionnel et le débat qui a eu lieu ici n'a levé aucune de nos craintes après le bac pro en 3 ans au lieu de 4 après la réduction de 30 % des enseignements généraux, avec l'augmentation désormais de 50 pour 100 des temps de stage, nous risquons d'arriver à l'os dans l'enseignement des disciplines générales et professionnelles, ces réformes sont le fruit d'un raisonnement utilitariste, selon lequel il faudrait répondre aux stricts besoins des employeurs, mais vous vous trompez car, y compris sur ce y compris sur ce qu'attend le monde de l'entreprise, dont les acteurs sont de plus en plus nombreux à alerter sur la nécessité d'apporter à nos jeunes, hein, au niveau de formation leur permettant d'évoluer tout au long de leur carrière, c'est aussi manqué cruellement d'ambition pour une jeunesse issus des milieux populaires concernant la revalorisation du métier d'enseignant, vous admettrez que nous sommes loin du choc d'attractivité nécessaire, premièrement parce qu'un tiers des crédits consacrés aux mesures de revalorisation ira à la mise en place du pacte enseignants c'est-à-dire conditionnée à la réalisation de missions certaines déjà pris en charge par les enseignants, ce qui n'a alors aucun sens, d'autres en regard de nouvelles missions, alors que nos enseignants travaillent déjà plus de 40 heures par semaine, ensuite parce que la promesse d'une revalorisation de 10 pour 100 de tous les enseignants concerne en réalité ne concerne en réalité que les enseignants de moins de 20 ans d'ancienneté, excluant de fait 2 tiers d'entre eux, le déclassement vécue par les enseignants et le résultat d'une très longue période de gel du point d'indice, bien difficile à rattraper aujourd'hui, résultat, même si des crédits sont sur la table, ils apparaissent bien loin de répondre aux enjeux et le personnel non enseignant est complètement oublié, à l'image des accompagnants d'élèves en situation de handicap quatre mille pardon recrutements prévus resteront trop peu nombreux au regard des besoins et qui continueront de vivre dans une extrême précarité défendre une école réellement inclusive implique de revaloriser ce métier essentiel par une meilleure rémunération par une formation renforcée, un statut qui les sortent de la précarité, enfin j'aimerais terminer en alertant sur l'inquiétude qui se développe dans les établissements scolaires, face à la hausse des coûts de l'énergie, l'Association des régions de France estime que le surcoût lié à l'inflation dépasse désormais les 200 millions d'euros pour 2022, et plus de la moitié des collèges, des lycées ne savent pas encore comment ils vont boucler leur budget d'ici la fin de l'année, de même, élus locaux et parents d'élèves s'interrogent en ce moment où l'on parle de délestage éventuelle du réseau électrique à dire, qu'adviendra-t-il des écoles si des coupures d'électricité doivent intervenir, nous avons besoin, Monsieur le Ministre, de réponse à cette question, les satisfecit que vous exprimez ne résiste pas à l'examen de ce budget, pourtant les dégâts causés par votre prédécesseur, nécessite de reconstruire des relations de confiance et une mobilisation générale au service des enfants et de la jeunesse, ce budget ne le permet malheureusement pas et nous ne donc nous ne le voterons pas. Merci, cher collègue, la parole est à madame Annick Billon pour le groupe Union centriste pour huit minutes. Monsieur le président, messieurs les Ministres, Madame et messieurs les rapports, les rapporteurs, monsieur le président de la commission, je souhaiterais commencer mon propos en saluant le travail de nos collègues rapporteurs, Gérard Longuet, Jacques Grosperrin et Nathalie Delattre depuis 5 ans, les crédits de la mission enseignement scolaire sont en hausse et ne nous nous ne pouvons que nous en féliciter, en juin, en 2023, le budget du ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse reste le 1er budget de l'État, cette trajectoire ascendante ne doit pas pour autant occulter des difficultés persistantes en cette rentrée, les étudiants ont subi les conséquences des 4000 postes non pourvus aux concours enseignants parmi les 12 millions d'élèves, certains se sont retrouvés sans professeur depuis plusieurs années pourtant, nous insistons sur le manque criant d'attractivité des métiers de l'enseignement avec mes collègues, Max Brisson et Marie-Pierre Monnier nous avons mené des travaux sur le bilan des mesures éducatives du quinquennat le constat est sans appel : seulement 4 % des professeurs des écoles considèrent que leur métier est valorisé est valorisé par la société, alors oui, Monsieur le Ministre, vous répondez en partie à ces écueils par des revalorisations salariales, devons nous nous en contenter non si elles sont absolument nécessaires, elles ne sont pas suffisantes, les enseignants devenir et néo-titulaires doivent pouvoir se projeter dans leur métier, ils doivent pouvoir y trouver un sens des perspectives de formation et d'évolution de carrière, ils doivent pouvoir y trouver où y retrouver l'envie d'exercer cette crise de l'attractivité frappe également la médecine scolaire en 2011 déjà, un rapport parlementaire suggéré d'améliorer le dispositif existant, 11 ans plus tard, un tiers des postes de médecins scolaires sont toujours vacants, avec en plus une forte disparité géographique Monsieur le Ministre, nous sommes face à un problème structurel qui s'enlise, d'année en année au par opportun de considérer les pistes présentées par la Cour des comptes en 2020, je souhaite également aborder le sujet crucial de l'éducation à la sexualité depuis plus de 20 ans, la loi impose l'organisation par les établissements scolaires pour tous les élèves du CP jusqu'à la terminal deux 3 séances d'éducation à la sexualité par an et par niveau ses obligations légales ne sont aujourd'hui pas respecté, seuls 10 % des établissements appliquent la loi et ce qu'qui mettent en place ces séances le font parfois sans recourir aux bons outils pédagogiques, elles sont donc pas peu ou mal dispenser, monsieur le ministre, avec mes collègues corapporteur de la délégation aux droits des femmes, Alexandra Borchio Fontan Laurence Cohen et Laurence Rossignol nous vous avons remis hier notre rapport porno l'enfer du décor, comme vous le savez le porno aujourd'hui est devenue pour nos jeunes, le lieu d'apprentissage de la sexualité par défaut, comme nous le disait cyniquement le professeur Israël Nisand nous n'éduquons pas nos enfants à la sexualité, rassurez-vous, la pornographie, le fait à notre place pour avoir échangé librement avec vous sur ce sujet hier, je connais votre volonté de faire appliquer la loi Monsieur le Ministre, nous partageons avec vous, l'ambition de bâtir une société plus égalitaire, sans violence, les cours d'éducation à la sexualité dès dès l'école primaire en sont une des clés et nous comptons sur votre détermination à les mettre en oeuvre sur l'ensemble du territoire et dans tous les établissements, comme le prévoit la loi simplement parlons aussi égalité la réforme du lycée, a provoqué une chute drastique des filles dans les filières scientifiques, les mathématiques doivent faire leur retour dans les programmes, et pas seulement à hauteur d'une heure et demie par semaine cette orientation stéréotypé se retrouve également dans l'enseignement agricole, monsieur le Ministre de l'Agriculture, les jeunes filles s'oriente principalement vers les cursus de services à la personne, alors que les formations dans le domaine de la production animale reste très masculine, parlons école inclusive l'école inclusive bénéficient de crédit en nette augmentation depuis plusieurs années, près de 4 milliards d'euros, ils seront désormais consacrer des efforts budgétaires substance substantielles ont été apportées au à ESH ces crédits à la hausse, la revalorisation des salaires des 132000 AESH et le déploiement des pial sont nécessaires en 10 ans le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés en classe ordinaire a connu une hausse de près de 60 pour 100 des effectifs dans le primaire et 150 dans le secondaire, ces efforts ne sont qu'une étape, les lacunes de la formation initiale et continue des AESH la faible rémunération persistante et les conditions d'exercice, nous oblige à faire évoluer leur métier pour eux et pour les enfants qu'ils accompagnent la proposition de loi en débat de la semaine prochaine, peut être un point de départ de plus, la multiplication des recrutements d'AESH 10 privé nous inquiète car elle entraîne une réelle rupture d'égalité l'enseignement scolaire ne se résume pas à l'éducation nationale, l'enseignement agricole mérite aussi toute notre attention, il est question de former des agriculteurs et des agricultrices pour demain, les effectifs en baisse et l'orientation souvent stéréotypés nous préoccupe l'attractivité de ces formations passe obligatoirement par une meilleure orientation par une orientation éclairé des outils existent, le camion du vivant, par exemple, mais sont-ils efficaces atteignent-t-il leur cibles j'en doute sur les aimé faire enfin je rejoins la position de la rapporteure, elles doivent pouvoir utiliser le plafond maximal prévu pour 2000 22 et 2023 compte tenu de la de la hausse des coûts de fonctionnement, les 10 millions d'euros, dont il est question, leur permettrait de pouvoir encaisser les hausses liées à l'inflation, permettez-moi, avant de conclure, de vous faire part d'un témoignage que j'ai eu pendant cette suspension puisque la discussion générale a eu a démarré tout à l'heure et nous nous sommes arrêtés, j'ai reçu à monsieur le ministre de l'Agriculture, un témoignage qui émane d'un directeur adjoint Jean François Vergnaud dans un lycée agricole de Vendée il me met il m'écrit cela et je voilà je j'espère qu'on aura des réponses à leur apporter nos jeunes enseignants embauchés en juillet ne sont toujours pas payés et ceux qui ont démissionné le sont toujours, cela illustre de gros dysfonctionnements du service RH du ministère de l'agriculture, donc j'espère qu'on trouvera des solutions au cours de cette soirée ou dans les jours qui viennent, pour répondre à ce cette problématique en conclusion, le groupe Union centriste votera unanimement les crédits de la mission enseignement scolaire mais sera vigilant sur les difficultés que je viens d'exprimer, je vous remercie. Dans la suite de la discussion, la parole est à madame Béatrice Gosselin pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président, messieurs les Ministres, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, après 2 ans de bouleversé par la crise sanitaire des craintes légitimes pesé sur le nombre d'enseignants présents dans nos dans nos classes à la rentrée 2022, comme cela a déjà été rappelé par mes collègues le budget de la mission enseignement scolaire connaît une forte progression de plus de six bien que 5 % avec 58 virgule 8 milliards d'euros hors pensions, auxquels il faut ajouter le fonds d'innovation pédagogique investir pour la France 2000 Tran 202032 150 millions d'euros malgré cette hausse, je souhaiterais m'attarder sur quelques points qui me paraissent importants et impacte le métier d'enseignant tout d'abord, la revalorisation des rémunérations des enseignants en début et en cours de carrière, on ne peut que se féliciter d'une rémunération de 2000 euros en début de carrière, mais pour poursuivre ses effets et rendre la profession plus attractive cette revalorisation doit se maintenir dans la durée et s'appliquer à l'ensemble de la profession afin d'avoir une cohérence dans la grille salariale, actuellement, le salaire médian de 2290 euros pour les enseignants est une rémunération assez peu élevé au regard du niveau de qualification et des 43 heures de travail hebdomadaire et mais à 1 135 milliards d'euros, la revue de l'harmonisation salariale envisagée répartis en une augmentation inconditionnel de 635 millions d'euros d'une et, d'une part, facultative de 300 millions d'euros pour les enseignants qui participeront au pacte à titre volontaire, mais les modalités de son pas de ce pacte sont peu précises et pas du tout évident à mettre en place, de plus, le déroulement de carrière reste lent et aléatoire,

Un 2ème point concerne les suppressions de postes prévues en 2023 depuis plusieurs années les l'éducation nationale les justifie par les projections démographiques liées à la baisse de la natalité, ce sont 2000 postes supprimés en 2023 pour une baisse démographique dans évalué à 92000 élèves, même si les inspecteurs d'académie, nous assure que le taux d'encadrement et de plus en plus élevée dans la Manche en compte cette année si celle enseignants pour 100 ton enfant à la rentrée de septembre pour les enfants du 1er degré j'entends, il n'en est pas moins que la suppression de poste fragilise les possibilités de remplacements de courte durée et impact la participation des enseignants à la formation continue, le 2ème point satisfaisant et la baisse du nombre de postes conjugué à une crise préoccupante du recrutement on constante, on constate, pardon, une tendance à la baisse des candidats au concours d'enseignement, avec 3700 postes non pourvus pour le concours de 2022, mais également une augmentation croissante des démissions dans la profession. On identifie plusieurs raisons à ce manque d'attractivité du métier d'enseignant en plus de la rémunération peu séduisante, on peut évoquer le manque de reconnaissance sociale des enseignants, le sentiment d'isolement et l'absence de soutien devant les difficultés. Les nouvelles conditions d'accès au concours externe avec des logiques différentes selon le cursus antérieur des lauréats semble complexe et pose le problème d'une charge de travail intense qui s'ajoute à la prise en responsabilité d'un groupe classe à temps plein ou à mi-temps selon les master, il est en outre indispensable que ces stagiaires soient accompagné par un tuteur au sein même de leur école dans les dans, là où il travaille, il faut également éviter les conditions d'exercice difficile pour un débutant classe unique poste partager entre plusieurs sites affectations dans des territoires peu attractifs, comme les REP devant des publics difficiles, les difficultés de recrutement entraînent de nombreuses disciplines en tension dans le second degré, notamment et l'absence de professeurs ou le défilé des remplaçants impacte fortement les chances de réussite des élèves depuis septembre, on déplore dans un lycée de l'ouest de la France, l'absence d'un professeur en terminale ST2S pour les cours de sciences et technologies de la santé et du social avec un coefficient 16 au Baccalauréat. Cette année, pour combler le manque d'enseignants, 20 % des postes étaient confiée à des contractuels et pour pallier le manque d'effectifs, la politique de recrutement largement relayée par la presse proposé 4 jours de formation avant une affectation ce métier exigeant ne s'apprend pas en 4 jours et les modalités de suivi de formation absolument nécessaires ne sont pas réellement explicité alors que la qualité de l'enseignement et de la pédagogie, d'un processeur sont des points essentiels pour la réussite des élèves, de de la le problème de mobilité des enseignants pardon les affectations après l'obtention du concours des néo-titulaires sont souvent éloignés du lieu de résidence, parfois même des contractuels renonce à passer le concours pour avoir la certitude de rester dans leur jeu, parlement se termine monsieur le et pour conclure, pour conclure, Amélie il faut améliorer l'attractivité du métier d'enseignant et cela suppose une cessèrent, revalorisation des salaires et une gestion plus humaine des ressources, je vous remercie.

Monsieur le président, messieurs les Ministres, Madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, D. R. et les crédits consacrés au remboursement de la dette qui deviennent, sous votre gouvernement, Monsieur le Ministre, le 1er budget de l'État, les crédits de la mission enseignement scolaire connaissent, il est vrai, une hausse de 6,5 mais peut-on s'en satisfaire, il est depuis longtemps reconnu que si notre pays figure en mauvaise position dans les classements internationaux, ce n'est pas par manque de moyens, mais par manque de réformes, la hausse des crédits doivent d'ailleurs être relativisée puisque 1 virgule 7 milliards correspondent à l'augmentation du point d'indice de la fonction publique et 400 millions à l'habituel glissement vieillesse technicité, une fois ces dépenses 1 virgule 9 milliards d'euros en année pleine doivent permettent de réaliser la promesse présidentielle d'un salaire des enseignants qui ne puisse être inférieure à 2000 euros cette remarque câble opération de communication ne vise cependant que les premières années d'exercice, la revalorisation en cours de carrière reste un mirage malgré que vous ayez à fermier, Monsieur le Ministre, que pour un professeur avec quelques années d'ancienneté l'augmentation pourrait aller jusqu'à 25 avant d'évoquer plus tard et plus prosaïquement un chiffre de 10 % or les 900 millions qui ont été inscrits à cette fin, ne correspondent pas réellement une augmentation mais seront liées à l'acceptation de nouvelles missions, dont la nature reste pour le moment très flou, il s'agit du fameux pacte l'attractivité de la profession souffre d'ailleurs de bien d'autres entraves j'évoquerai les conditions de travail dégradées, une insécurité grandissante, une absence de reconnaissance, une perte d'attractivité des perspectives de carrière limitée et aléatoire, un temps de travail important comprenant la part invisible des corrections de devoirs et des tâches administratives et des affectations territorial, aléatoire qui rendent difficile la conciliation entre vie professionnelle et vie privée à cela, le gouvernement n'apporte aucune réponse 3000 750000 postes d'enseignants sont non pourvus cette année et à ce chiffre à ce chiffre a triplé entre 2021 et 2022 les concours ne font pas le plein de candidats, les démissions se multiplient, surtout si les jeunes enseignants dont nous dénonçons depuis des années leur affectation systématique aux postes les plus difficiles, pourtant, vous avez décidé de supprimer 2000 postes d'enseignants pour suivre l'évolution démographique, où est la logique de tout cela, les enseignants font part de leur découragement face au manque de soutien de la part du ministère, les récentes polémiques sur la défense du principe de la laïcité sont révélatrices d'un profond malaise en raison de l'absence de ligne claire du gouvernement en peine à distinguer une feuille de route pour les prochaines années, je ne reviendrai pas sur tous les points développés les questions présenté par Jacques Grosperrin et Max Brisson nos excellents collègues car pour ma part, je prendrai l'exemple du sujet qui m'est cher, celui du sport à l'école, convaincu de l'importance du sport pour la santé et pour l'équilibre de nos jeunes, je déplore le manque manifeste de moyens et d'organisation permettant de mettre en place les 30 minutes d'activité physique à l'école, qui sont, je le rappelle obligatoire ah sont qu'entre 10 et 20 % par les chefs d'établissement je m'interroge donc sur la volonté gouvernementale de rendre effective cette mesure de santé publique, je poserai la même question concernant les mesures à prendre pour le savoir nager, de nombreux enfants ne découvrent la natation comme moyen des cours dispensés par l'école, or l'accès au cours semble très aléatoire, sans que nous puissions avoir une vision d'ensemble, selon les années et les établissements au moment où la crise de l'énergie va venir compliquer encore davantage l'organisation de ces cours en mettant en péril l'ouverture des piscines, quelles actions envisagez-vous, Monsieur le Ministre, pour garantir l'effectivité de cet apprentissage, qui est essentiel, aussi bien sur le plan de la sécurité que de l'activité physique dans ce domaine comme dans bien d'autres, les annonces sont là, mais à peine à trouver leur traduction dans des actes, je pense que l'éducation nationale mérite mieux que des mesures d'affichage et pour conclure sur ce budget je le redis, si l'éducation a bien besoin de moyens à la surtout besoin de vraies réformes

Monsieur le le président, messieurs les présidents de la commission des finances et de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, monsieur le rapporteur spécial madame et monsieur les rapporteurs pour avis, mesdames et messieurs les sénateurs. Avant d'aborder les crédits de la mission enseignement scolaire je voudrais d'abord vous remercier pour la qualité des échanges que nous avons eu depuis plusieurs mois les débats en commission comme la lecture des rapports que produit le Sénat sont autant d'apport essentiel dans nos réflexions et dans l'élaboration de nos politiques publiques permettez-moi aussi d'exprimer l'honneur et le plaisir qui sont les miens au moment de présenter le budget de l'école pour 2023, dans un contexte de croissance continue depuis 2017, ce projet de loi de finances, marque une rupture dans l'ampleur de l'effort budgétaire proposée et dans les ambitions transformatrices qui sont associés, je suis convaincu que nous nous ils sont ainsi au niveau des attentes qui sont légitimement exprimer vis-à-vis de l'école à ce sujet, et avant d'entrer dans le détail des axes de ce budget, je voudrais revenir sur le travail réalisé depuis 6 mois, puisque certains d'entre vous ont questionné mon volontarisme. Le projet de loi de finances pour 2023 propose ainsi un budget à 59,7 milliards d'euros pour l'éducation nationale en croissance de 6,5 pour 100 par rapport à 2022 autour de plusieurs axes prioritaires premièrement, et la première de ses priorités, c'est bien entendu la revalorisation des enseignants, l'amélioration de l'attractivité du métier enseignant est un défi majeur, l'enjeu est loin d'être uniquement français, du reste, comme votre rapport l'a récemment souligné monsieur le rapporteur longue néanmoins la France un un effort particulier à faire pour améliorer les salaires de ses professeurs, notamment en début et en milieu de carrière comme le recommande votre rapport cet effort nécessaire que vous appelez de vos voeux, nous le faisons dans ce budget, il y a un niveau inédit, la revalorisation des enseignants représentent une enveloppe totale de 1 135 milliards d'euros pour 2023, un montant qui couvre les 4 derniers mois de de 2023 la revalorisation entrant en vigueur en septembre, l'effort sera donc amplifié en année pleine des 2 1000 24 je ne reviendrai pas ici en détail sur les 2 volets de cette revalorisation une part socle qui permettra de rehausser en moyenne de 10 % les enseignants, avec une priorité donnée à la première moitié de carrière et un pacte associé à des missions nouvelles et à des missions mieux reconnu en bref un dispositif porteur à la fois d'un regain d'activité des carrières et de transformation de notre école, cet effort considérable qui concernera l'ensemble des enseignants est à la hauteur de la place que les professeurs occupent et doivent occuper au coeur de la cité, plus que jamais, en effet, nous devons réaffirmer l'importance cruciale des enseignants dans notre pays le respect qui leur est dû, doit aller de Pair avec une meilleure reconnaissance financière par par leur employeur, l'État et c'est ce que nous faisons avec ce budget, mais, et je sais que c'est la préoccupation de vous toutes et tous, l'attractivité du métier d'enseignant ne se résume pas à un niveau de rémunération, c'est aussi de sens de reconnaissance de soutien que les professeurs en particulier les plus jeunes ont besoin, c'est un chantier complexe pour lequel nous nous inspirons des recommandations de votre rapport, monsieur le sénateur. Aller vers davantage de travail collaboratif mieux accompagner les professeurs débutants voici par exemple des axes qui nous paraissent pertinents et qui nourrissent nos projets pour 2023, nous travaillons également sur la gestion des ressources humaines sur les déroulé de carrière pour mieux répondre aux attentes des enseignants, en particulier les plus jeunes, cet effort de revalorisation concernera aussi les autres professionnels de l'éducation nationale pour un montant de 140 millions d'euros, en particulier nos médecins et infirmiers qui joue un rôle central pour la santé et le bien-être de nos élèves bénéficieront pour les 4 mois de 2023 d'une enveloppe de 6 8 millions d'euros, la 2ème, priorité de ce budget, c'est la réussite de tous les élèves cette priorité nous est commune, j'ai pu le constater au travers des amendements que vous avez déposé, déposé, nous allons tout d'abord améliorer le taux d'encadrement grâce à la volonté du gouvernement de ne pas répercuter directement la baisse démographique à venir sur le nombre d'enseignants, nous aurons 100000 élèves presse à peine 100000 élèves de moins à la rentrée 2023 par rapport à la rentrée 2022, c'est considérable, et cela va durer tout au long du quinquennat en contenant la baisse du nombre d'enseignants, nous continuons à améliorer le taux d'encadrement en primaire et nous le maintenons dans le secondaire, en second lieu nous amplifions les dispositifs en faveur de la réussite des élèves tels que les dédoublements en REP, plus le plafonnement à 24 des classes de primaire aurait et le développement des classes Ulis la réussite des élèves passera aussi et surtout par des réformes structurantes comme celle des lycées professionnels que nous portons avec la ministre, Carole Granjean et qui fait actuellement l'objet d'une concertation bien engagée, j'ai déjà évoqué l'importance du collège, sur lequel un travail de transformation s'engage au bénéfice de la réussite de tous les élèves le 3ème point c'est mon souhait, à travers ce budget de donner corps à la priorité que j'ai fixé en matière de lutte contre les inégalités, nous serons plus attentifs que jamais aux plus fragiles pour que chaque enfant, chaque jeune dans tous les territoires puissent suivre sa scolarité dans les meilleures conditions de nombreux dispositifs petits déjeuners gratuits, contrats locaux d'accompagnement territoire éducatif ruraux seront étendues grâce à des à des crédits supplémentaires, les bourses de collège et de lycée ont été revalorisés à la rentrée de 4 % et nous nous fixons également des objectifs ambitieux de meilleure utilisation des fonds sociaux disponibles dans les établissements, il faut que toutes les familles qui en ont besoin puissent avoir accès à ces aides sur ce sujet, un amendement du gouvernement visant à abonder les fonds sociaux des établissements d'enseignement agricole a été déposée, il permettra en toute cohérence, d'aider l'ensemble des jeunes qui en a besoin, quel que soit leur établissement sur ce sujet comme sur les autres amendements qui concerne l'enseignement agricole, mon collègue ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, que je remercie pour sa présence pourra apporter toutes les réponses nécessaires, les enjeux de l'enseignement agricole sont en effet majeur pour la formation de nos jeunes et pour l'avenir de notre pays, le 4ème point ce c'est le le fonds d'innovation pédagogique qui sera doté pour l'année 2023 de 150 millions d'euros et ce fonds est une vraie nouveauté, il va permettre de financer tous les projets pédagogiques innovants portés par les équipes éducatives qui seront issus des débats engagés dans le cadre du Conseil national de la refondation en nous fondant sur l'expérience conduite à Marseille, nous préparons le déploiement d'un dispositif ambitieux dans son volume novateur dans son fonctionnement, puisqu'il sera pleinement pleinement déconcentré est ainsi proche du terrain, je ne doute pas que cette approche concrète local recueille l'approbation de votre assemblée, ce nouveau fonds qui viendra abonder notre budget à partir d'un transfert de crédits de la mission investir pour la France 2030 permettra par exemple de financer des projets autour des savoirs fondamentaux de l'inclusion des élèves en situation de handicap de l'éducation artistique et culturelle, le tout sans mise en concurrence et dans un esprit de confiance faite aux équipes pédagogiques afin de faciliter le financement de ces projets, en particulier dans le 1er degré, je soutiendrai l'amendement que vous avez déposé, monsieur le rapporteur Grosperrin votre texte constitue une mesure de simplification efficace et je ne peux qu'y être favorable, pour terminer, je veux revenir en quelques mots sur un sujet important sur lesquels je sais que vous êtes impliqué, celui de l'école inclusive qui demeure plus que jamais une priorité 4000 nouveaux postes d'AESH seront créés à la rentrée 2023, après une hausse identique en 2022, les moyens sont là, cette hausse continue doit s'inscrire dans le cadre d'une réforme plus globale, celle de l'acte de de l'école inclusive, l'objectif de la réforme venir est simple et ambitieux que chaque enfant soient correctement accompagnés en fonction de ses besoins, nous avons engagé le travail avec un cap très clair : présenter des propositions concrètes lors de la conférence nationale du du handicap, qui aura lieu au printemps 2023, il s'agira notamment de définir les modalités permettant aux AESH d'atteindre, si c'est leur choix, un temps plein de trente-cinq heures conformément à l'engagement du président de la République, afin d'améliorer immédiatement la situation financière fragile des ESH les avais sages vont devenir éligibles aux primes Rep et Rep plus comme les à ED et connaîtront en outre une revalorisation globale de 10 % en septembre prochain, mesdames et messieurs les sénateurs, vous le voyez, ce budget est ambitieux et répond à des constats que nous partageons très largement, j'en suis convaincu, je vous remercie. nous allons passer à l'examen des amendements à l'article 27 à l'état B, nous allons commencer par le 916 madame de Marco. Merci monsieur le président, donc je l'ai déjà dit en discussion générale, le constat est déjà établie en encore ans les enseignants ont subi une perte de pouvoir d'achat massive les rapports Regards sur l'éducation publié par l'OCDE appuie largement ces chiffres puisqu'ils estiment qu'entre 2000 et 2019 alors que les salaires des enseignants a augmenté dans la plupart des pays de l'OCDE, c'est en France que le salaire le plus diminuer avec une baisse qui atteint 10 % dans l'enseignement secondaire, toujours selon l'OCDE, le salaire statutaire des enseignants du primaire et du secondaire a pris 10 ou 15 ans de service est inférieur d'au moins 15 % à la moyenne de l'OCDE, cette situation du décrochage des salaires, l'une des raisons majeures du déficit de recrutement de la profession, bien qu'elle ne soit pas la seule, or les moyens alloués dans le budget 2023 ne nous semble pas à la hauteur de l'enjeu, tout d'abord l'enveloppe ne répond pas à la promesse initiale du président de la République de revaloriser inconditionnellement les salaires des enseignants de 10 la part conditionnel 300 millions d'euros entre septembre et décembre 2023 correspond en réalité à des tâches déjà effectué par les équipes pédagogiques, le rapport de juin 2022 notre collègue et rapporteur Gérard Longuet vingt dans le même sens et conclut lui aussi à les différences salariales entre la France et d'autres pays, son nom corrélés autant de service des enseignants français nous considérons donc que l'augmentation inconditionnel de 10 pour 100 des enseignants et de droit au regard du décrochage de leur salaire et de leur engagement sans faille pendant la crise sanitaire, par ailleurs, nous considérons que tous les enseignants doivent être augmentés, quelle que soit leur ancienneté selon nos calculs et ceux des syndicats, il faudrait ainsi plus d'un milliard d'euros supplémentaires en année pleine, par rapport à ce qui était proposé, voilà, c'est précisément le but de cet amendement. Chers collègues en discussion commune 888 madame Monnier. Merci monsieur le président, donc, les arguments sont un peu les mêmes simplement le montant est supérieur à celui proposé je reprendrai quand même un élément le des cons accrochage est vraiment paradoxal parce que comment expliquer que la rémunération ne professeur des écoles recrutés à bac plus cinq sont aujourd'hui inférieurs au salaire moyen des fonctionnaires de catégorie B, c'est quand même quelque chose qui est grave dans ma des j'ai j'ai expliqué qu'on allait arriver un effet de plateau et qu'on ne prenait pas en considération ce qu'il avait plus de 20 ans d'exercice et que, finalement, à l'heure où ce budget prévoit d'allouer le même montant de 300 millions pacte enseignants qui conditionne pour sa part, l'augmentation de salaire au fait d'assurer de nouvelles missions pour nous, c'est un choix politique autre auquel nous ne souscrivons pas. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Ici des finances monsieur le président, est défavorable à ces deux amendements non pas qu'il soit antipathique mais il viderait de leur sens le programme vide la qui serait amputé des trois-quarts de de ses recettes et le programme soutien du ministère qui serait amputé sans doute de plus de de près de la moitié est donc défavorable. Merci, monsieur le Ministre.

or le gouvernement porte déjà une mesure inédite de revalorisation des enseignants qui représente 1 virgule 9 milliards d'euros dans sa part inconditionnel en année pleine, à quoi s'ajoute une part conditionnel à à hauteur de 300 millions d'euros pour les 4 derniers mois de l'année 2023 cet effort aura des effets tangibles puisque l'entrée dans la carrière ne se fera pas à moins de deux mille euros et cela sera garantie, avec une hausse totale que nous proposons, qui pourra, avec l'acceptation des missions supplémentaires atteindre 20 % voire en effet 25 % pour de jeunes enseignants adhérent au pacte et donc pour toutes ces raisons et parce que nous portons déjà une mesure ambitieuse de revalorisation des professeurs, j'émets un avis défavorable à vos amendements. Merci, monsieur le Ministre, dont je les maisons voile et tout d'abord le 916 avec 2 avis défavorables. C'est pour qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté même vote pour 888 même vote il n'est pas adopté. Parce qu'on a 2 amendements discussion commune de 866 Monsieur Bresson. Oui, merci Monsieur le Président, cet amendement d'entrée Richard et de 47 sénatrices et sénateurs concerne les AESH dont nous allons beaucoup parler ce soir et c'est justice puisqu'on connaît la difficulté de leur tâche et la précarité institutionnelle de leur situation aujourd'hui, leur nombre était insuffisant pour répondre aux modifications des BD des BD MDPH, résultat d'un département à l'autre, la prise en charge est différente, ce qui n'est pas acceptable là les réponses collectives ou personnalisés sont si arbitré par les pial sans prise en compte réelle de la notification de la haine cet amendement vise donc encourageait le gouvernement a augmenté de 10 % le nombre des avait sage, il propose d'investir de 134 millions en faveur de l'inclusion scolaire, cela ne réglera certes ni la faiblesse de rémunération, ni l'absence de formation des AESH cet amendement comme beaucoup d'autres, ce soir, ce sont des signaux d'alerte l'école inclusive ne se fera donc pas sans une politique globale de prise en charge de l'enfant en situation de handicap dans le temps de l'école qui ne se résume pas autant de classe, vous propose une bouffée d'oxygène qui serait la bienvenue, vous venez de parler Monsieur le Ministre de l'acte de de l'école, cuisine, mais nous vous êtes pas dans votre discours est dans une logique partenariale avec les autres acteurs qui seul réglera la prise en charge globale des enfants en situation de handicap tout au long de la journée d'école avant, pendant et après la classe. Merci le 887 madame Meunier. Merci monsieur le président, les retours de terrain sont très clairs, ils indiquent que l'éducation nationale prend plus ou moins en compte les notifications MDPH notamment faute d'AESH nombre insuffisant Max Brisson, vient de parler de situation différent complètement différente, c'est vrai, d'un département à l'autre, moi, je cite. Sur la Seine-Saint-Denis 2500 enfants qui ont une notification sans, sans, à ESH, c'est quand même un chiffre qui est impressionnant, passe par ailleurs, c'est que certaines familles en arrive à rechercher par elle-même des solutions ou par le biais d'associations des des AESH 10 privé et, selon les associations de parents il y a un marché de l'accompagnement privé qui est en train de se développer, même s'il est encore difficilement quantifiables, je trouve cette privatisation de l'accompagnement du handicap, est très inquiétante et ça provoque vraiment une rupture d'égalité et rend renforce les inégalités sociales. Président, mes chers collègues, ces ces deux amendements sont inspirés par une préoccupation qui est légitime et qui force, celle des familles. Les la commission des finances, a émis un avis défavorable, mais je voudrais faire une remarque un peu plus de, de, de, et interroger Monsieur le Ministre, l'inclusion est une responsabilité nationale. Qui relève donc de la solidarité. L'éducation nationale doit-il être le seul ministère en charge de ceux-là, c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Je vous rappelle que les MDPH sont comme leur nom l'indique départemental. Et quel prescrivent les le statut d'AESH et l'attribution d'AESH sans qu'il n'y ait de véritables concertations avec l'éducation nationale, qui a des capacités spécifiques ou qui est en mesure d'évaluer la situation de chaque élève, encore que Monsieur le Ministre, reconnaissons que ce qui manque parfois à l'éducation nationale et surtout dans les grands établissements, c'est un lien entre entre l'établissement et l'élève handicapé quand les établissements sont plus petits, force des reconnaissent qu'ils sont peut-être moins rationnel, mais au moins il y a ce lien et on peut évaluer la situation de l'enfant qui est, qui est, pour lequel la MDPH demande une prescription d'AESH je souhaite profondément que l'on est un travail interministériel et avec l'ADF sur ce sujet parce que sinon, on est dans une situation que je qualifierai de fuite, c'est-à-dire quand il y a un problème à la MDPH on renvoie la responsabilité au ministère qui lui doit s'occuper de tous les élèves et tous les enseignants et dont les moyens sont quand même. Ne sont pas illimitées, je rappelle que ces deux amendements l'amendement d'André Richard et que dont je comprends très bien le à lui seul représente la moitié de la mission du programme, soutien de l'éducation nationale, ça veut dire que pouf le ministère perd la moitié de ses moyens, votre amendement était plus raisonnable, madame en terme de prix de coûtent plus exactement, mais il s'applique sur le programme, soutien de l'élève de mémoire et représente une ponction considérable sur ce programme, ce qui veut dire que ce sont je l'estime profondément des des amendements d'appel, monsieur le Ministre, vous avez la responsabilité, vous appartenez un gouvernement vous n'êtes pas seuls dans ce gouvernement, je crois qu'il faut que vous puissiez rassurer au plus tôt le Parlement parce que vous aurez la même question à l'Assemblée nationale en en montrant qu'il y aura un fardeau partagé, mais aujourd'hui ce serait. Injuste de faire peser sur la vie de l'élève, d'une part, et sur les moyens du ministère, d'autre part, une responsabilité qui doit être maîtrisée, contrôlé, ce qui suppose un peu définition et ensuite partagée entre les différentes sources de solidarité et le ministère de l'éducation n'est pas la seule. Merci, monsieur le Ministre. Merci monsieur le Président, Madame, Monsieur le Sénateur, madame la sénatrice, nous avons créé 8000 postes d'AESH en 2000 24000 postes en 2021, 4000 en 2022 ici, vous approuvez ce budget 4000 en 2023 pour un total qui dépasse les 130000 postes d'AESH, c'est le 2ème métier de l'éducation nationale pour vous donner une idée de ce que ça représente et en effet, nous avons des des difficultés à répondre aux notifications qui viennent de façon très très insistante et et c'est légitime, bien entendu de la part des MDPH, par conséquent, il ne s'agit pas simplement de, de, de créer des postes d'AESH c'est ce que nous faisons, il faut aussi repenser plus structurellement les conditions d'accueil des élèves en situation de handicap et c'est précisément ce qui est en train de se préparer en vue de la conférence nationale sur le handicap, qui aura lieu au printemps un comité interministériel a été mis en place, nous allons échanger avec les collectivités, en particulier les départements, une réunion est prévue à ce sujet le 15 décembre et nous travaillons de manière à également avec les MDPH de manière à mettre à plat le système pour parvenir à cette conférence nationale sur le handicap, les progrès sur l'école inclusive, c'est pour cela que j'ai parlé d'acte de de l'école inclusive ne peuvent pas simplement être remplies par les postes d'AESH et leur multiplication, mais par une réflexion plus globale et plus structurelles sur l'accueil des enfants en situation de handicap, de manière à le pérenniser dans le temps d'un point de vue budgétaire également pour l'éducation nationale et pour les meilleures conditions d'accueil des enfants concernés et donc pour ces raisons, j'émets un avis défavorable à ces amendements.

on a du mal à trouver des personnels et puis la manière dont la prise en charge des enfants en situation d'être dans le handicap s'effectue et relativement fragmenté sur le terrain, ce qu'il appelle sans doute Monsieur le Ministre des réflexions pour savoir s'il ne serait pas opportun d'envisager, en la matière une décentralisation de de la responsabilité des AESH parce que finalement, il serait cohérent qu'il puisse y avoir la la décision par la MDPH et la prise en charge, pourquoi pas, par les départements, en tout cas, cela permettrait sans doute d'avoir une meilleure prise en charge de l'ensemble de la des enfants en situation de handicap et puis aussi de rapprocher la décision du terrain, je pense qu'une réflexion doit se de s'initier là dessus. Merci, cher collègue, madame la présidente Gruny. Oui merci monsieur le président, monsieur le ministre, je vous ai écouté attentivement, vous avez dit qu'il fallait réfléchir simplement on réfléchit pendant combien de temps parce que nous, ce qu'on a sur sur le terrain, ce sont des parents désemparés, des gamins perdus, moi je suis dans le département de Len 1er département pour l'illettrisme, l'année prochaine on va inaugurer la Cité de la francophonie c'est le berceau de la langue française, on est complètement oublié des aveux SH, on en a besoin, mais on a besoin aussi d'AESH, formé, c'est-à-dire le nombre formés rémunérés parce que le métier n'est pas attractif aussi parce que ne permet pas de vivre décemment, donc réfléchir, on est tout à fait d'accord, on veut bien vous aider, moi je travaille avec le directeur académique la MDPH je suis conseillère départementale mais sincèrement, on en a assez de réfléchir, donc quand est-ce qu'on aura fini cette réflexion merci. Merci madame Meunier. merci Monsieur le Président, c'est vrai que le vote a été fait d'une école inclusive et de faire des pial et que dans donc ouvrir l'école à l'enceinte des enfants handicapés parfois ses enfants auraient besoin d'aller dans d'autres structures comme des Ulis ou dixième, malheureusement, le nombre de places en est restreint et cela fait donc que l'école doit apporter une réponse à des enfants avec un accompagnement qui n'est pas à la hauteur, donc ça il faut l'intégrer aussi dans la réflexion que vous allez avoir et puis je crois que vous voulez arriver à 100 % de de couvertures et qu'il faudrait prévoir une augmentation de 12,6 % des postes pour s'approcher de ce Tour de couverture, ça voudrait dire qu'il faudrait prévoir 10270 postes supplémentaires pour 2023 et pas 4000 même si c'est un effort qui a été fait, ce n'est pas suffisant pour arriverait à vraiment avoir une couverture efficace. Si Monsieur Bresson. Bresson. Je ministre c'est vrai que depuis le la loi pour une école de la confiance des progrès ont été réalisés et ce serait pas pas juste de ne pas l'indiquer et de de pas le dire, la situation était encore beaucoup plus médiocre avant la loi portée par Jean-Michel Blanquer, mais pour autant, l'école inclusive n'est pas au rendez-vous, elle n'est pas à la hauteur de cette belle mission que l'école voudrait se donner et je crois que sur le sujet, il nous faut tous faire preuve de grande modestie, parce que de toute la France le recul le retard a été largement accumulées au cours des années, la réponse ne peut pas être que quantitative, mais vous comprenez, ici, que tout au long de la soirée, on va mettre en avant la précarité institutionnelle que les AESH subissent et qui êtes indignes dans un grand pays comme le notre, le notre, notre rapporteur spécial ah je crois poser le vrai sujet, celui de la manière dont on aborde une politique globale et partenariale de la prise en charge de l'enfant en situation de handicap, la réflexion sur le chef de file à épouser et on peut se c'était rouge et d'ailleurs sur le ce, pour savoir si l'éducation nationale est le mieux placé pour assurer ce chef de file à compte tenu de ce que sont ses ses compétences, sa culture et ça m'a, hier, d'être organisée en tout cas, la question se pose, et c'est comme cela qu'il faut aborder les concertations dont vous nous avez parlé donc je rejoins la proposition de Gérard Longuet, l'absence d'articulation est une vraie faiblesse de même bien sûr que l'hétérogénéité des situations d'un département à l'autre, qui pour le Girondin que je suis, excusez-moi, monsieur le Ministre, n'est pas acceptable et nécessite un cadrage national interministériel comme vous l'a proposé le Gérard Longuet je retirerai l'amendement d'André Richard, à la suite des la demande du rapporteur. Merci donc, le 866 s'est retiré du jeu, je fais voter sur le 887 avec 2 avis défavorables. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté cet amendement discussion commune 914 Madame de Marco. Oui merci la situation des AESH n'est pas acceptable, nous le disons, ce constat est vraiment partagée sur tous les bancs qu'moins accepter que cette profession féminine à 90 % vivent largement en dessous du seuil de pauvreté, que leur rémunération moyenne s'établissent à 850 euros Net comme accepter qu'une telle fonction pourtant vital au sein de l'école dite inclusive soient rémunérés de manière aussi indigne, c'est pourquoi nous vous proposons, très simplement, d'augmenter de 10 % l'enveloppe budgétaire dit dédié à la rémunération des AESH cela ne doit être qu'un début, un 1er pas qui devrait être ensuite poursuivi avec un objectif simple : aucune AESH en dessous du SMIG. Merci monsieur le président, sans 32000 ASH et 93 % de femmes qui jouent un rôle fondamental dans le cas de l'école inclusive pour assurer la scolarisation des élèves en situation de handicap dans les meilleures conditions, ces personnels ne bénéficie pourtant pas de la reconnaissance qu'il mérite et font face à une grande précarité, ils font parfois même pas partir ou ne sont pas considérés comme faisant partie de l'équipe éducative, ils sont parfois sur plusieurs établissements avec un emploi du temps qui changent très rapidement avec des différences aussi de traitement au sein des départements, il y a vraiment besoin d'une harmonisation contrainte de travailler à temps incomplet, la majorité d'entre eux bénéficient d'une rémunération extrêmement faible hein moyenne de une moyenne de 850 euros par mois exerce dans des conditions très difficiles, aggravées dans la période récente, par la mise par la mise en place des pieds à l'affectation auprès de plusieurs enfants, parce que maintenant il y a beaucoup plus de mutualisation, plutôt qu'une aide individualisée au sein de de différents et multiplication des déplacements avec monsieur le ministre, une vraie question sur le remboursement des frais de déplacement et un changement vraiment très fréquente de leur emploi du temps, alors c'est vrai qu'il a eu 80 millions d'euros qui ont été intégré par le gouvernement au présent PLF suite au 49 3 c'est un 1er pas mais la marche est encore haute pour garantir une rémunération décente. Ne serait-ce que pour atteindre le seuil de pauvreté parce que, même avec l'augmentation que vous prévoyez, il sera encore en dessous du seuil de profs pauvreté c'est pour soi que nous proposons d'abonder le fonds de 20 millions d'euros supplémentaires, et j'en profite pour interroger le ministre-sur les modalités de répartition de cette enveloppe de 80 millions d'euros permettra-t-elle réellement d'augmenter l'enceinte des ASH de plus de 10 % ou bien est-ce que cette augmentation sera conditionnée par l'acceptation de nouvelles missions, notamment durant le temps périscolaire

aujourd'hui, on assiste à un turn-over assez importants dans ce métier parce que évidemment les femmes puisque ce sont souvent des femmes qui exercent cette profession quand elle trouve quelque chose de plus rémunérateurs, s'en va. S'en vont, pardon, or il y a un enjeu de professionnalisation et on a besoin donc de fidéliser dans ces métiers et ça passe par d'importantes revalorisations est, en effet, Monsieur le Ministre, que vous venez de rappeler, c'est-à-dire les 10 % d'augmentation en septembre prochain, comme les primes plus ne permettront pas à ses salariés d'être au-dessus du seuil de pauvreté, et vous venez vous-même de dire que ah ESH c'est le 2ème métier de l'éducation nationale, je pense que ça n'est pas tolérable que dans un pays comme la France le 2ème métier de l'éducation nationale soit rémunéré en en dessous du seuil de pauvreté, et enfin pour apporter notre Pierre au débat qui s'est engagé et qui me semble tout à fait intéressant sur comment on conçoit l'accompagnement des enfants dans l'ensemble de leurs vies d'enfants, pas seulement d'ailleurs la scolarité, il me semble que le statut de la fonction publique est un qu'il faudrait travailler parce qu'il est intéressant parce qu'il permet, notamment, des passerelles entre la fonction publique territoriale et la fonction publique nationale d'état et que, il y aurait des choses à imaginer pour que précisément ce nouveau métier d'AESH accompagnants des enfants soit encadré dans un statut de la fonction publique territoriale, avec toutes les passerelles entre collectivités éducation nationale. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le droit à l'éducation pour tous les enfants en situation de handicap est un droit fondamental que le président de la République a placé parmi ses priorités pour ce nouveau mandat l'école inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la maternelle au lycée, par la prise en compte de leur singularité, de leurs besoins éducatifs cet amendement d'appel vise à encourager le gouvernement à revaloriser l'ensemble des rémunérations des AESH à les encourager à employer leur droit à la formation et à la validation des acquis de l'expérience et à leur proposer davantage de contrats à temps plein, le mécanisme est un peu plus modeste que les précédents, mais le le but est le même, merci. Merci le 483 identique, madame la présidente de l'autre. Oui, il est défendu le but était de dire que le RDSE s'associer à ce combat sur les AESH, merci. Merci de 595 Mabillon. Oui, merci Monsieur le Président, on est toujours sur les AESH ASH il est-il proposé avec cet amendement, d'attribuer 5 millions d'euros supplémentaires en faveur de de l'action 03 inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, donc d'autres amendements ont proposé des enveloppes différentes donc cette enveloppe de 5 millions me semble assez raisonnable à l'écoute de tout ce que j'ai pu entendre jusqu'alors, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit que je partage bien entendu sur ces bancs sur le métier, SH. Merci de 898 n'est pas défendu, il tombe, monsieur le rapporteur sur les 6 amendements en discussion commune. Monsieur le président, le le premier amendement 914 est un amendement significatif pour la commission des finances par le la somme qu'il se propose de d'ajouter : ce n'est pas un un, un amendement d'appel, c'est 5 % d'augmentation c'est simplement pas possible à financer puisqu'on est encore dans le pré, les dans le un prélèvement significatif sur la vie de l'élève qui n'est, qui correspond à un véritable besoin dans les établissements, nous le savons les uns et les autres sur l'ensemble des amendements d'appel la commission des finances souhaitent le retrait tout en en comprenant là l'opportunité et la pertinence, les indications que monsieur le ministre nous a donné, et en particulier ce contact permanent avec les associer à les grandes associations nationales d'élus locaux. Me paraît de bon augure et et permet de répondre un petit peu à mon excellente collègue Pascale Gruny il faut faire quelque chose, mais on ne fait pas rien je dirais de majorité en majorité cette prise en charge de de l'enfance handicapée dans une école inclusive a considérablement progressé et reconnaissant qu'il y a une telle diversité, c'est la raison pour laquelle quand vous évoquez le statut de la fonction publique territoriale oui naturellement, mais il y a une telle diversité d'handicap et une diversité dans les les besoins que les les les enfants handicapés exprime sur le chemin ou d'une inclusion d'une intégration ou d'une intégration marginal qu'il est extraordinairement difficile d'avoir un standard absolu, c'est la raison pour laquelle, pardonnez-moi, je suis un peu long mais on a vraiment besoin d'avoir entre les responsabilités ministérielles et locales, des, des critères d'actions qui soit beaucoup plus, enfin, la prescription obligatoire qui n'est pas discuter, qui n'est pas évalué, qui n'est pas établi abouti et nous sommes à la commission des finances, gardien des finances publiques un un facteur de d'inconnus qui ne permet pas de mettre l'argent nécessaire là où il faudrait le mettre, si on a entre pas dans le détail et ce détail aujourd'hui n'est pas maîtrisé cette organisation pratique n'est pas maîtrisé et je pense qu'il faut aller, on a une belle somme, déjà on peut faire mieux, on peut faire mieux, mais il faut savoir comment et on ne le sait pas, ça c'est à cet instant. Merci, monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, le gouvernement partage mesdames et messieurs les sénateurs, votre préoccupation d'augmenter la rémunération des ESH cela se fait d'abord par des primes en éducation prioritaire pour les AESH, comme pour les ED qui seront versées à partir de la rentrée 2023, cela se fait aussi par une augmentation inconditionnel de 10 pour 100, et nous avons retenu en première lecture un amendement de l'Assemblée nationale pour cela une augmentation de 10 pour 100 inconditionnelle pour tous les AESH à la rentrée 2023, mais au-delà de ces avancées, je mentionnerait aussi l'effort de de formation des avait sache qui accompagne ce mouvement au-delà de cela, ce qui est nécessaire, c'est d'augmenter le temps de travail des avait sage car leur faible rémunération est lié à un temps de travail hebdomadaire trop faible d'environ 24 heures nous devons ton donc tendre vers les 35 heures, et pour cela, nous travaillons avec les collectivités dans la perspective de la conférence nationale sur le handicap pour s'engager dans l'acte de de l'école inclusive, de manière à ce que les AESH soit payé à hauteur des tâches qu'ils accomplissent et soit payé également à hauteur d'un volume hebdomadaire horaires qui leur permettent, bien entendu, de toucher des rémunérations satisfaisantes, c'est pourquoi j'émets un avis défavorable à votre amendement à vos amendements, tout en partageant bien entendu l'ambition qui est celle de mieux rémunérer nous avait sache cette ambition se traduira dès la rentrée, mais elle devra prendre tout son sens dans le cadre de la conférence nationale pour le handicap.

conviendrez que c'est un drôle de métier dont on ne peut pas vivre correctement et un drôle de métier si peu attractif en termes de reconnaissance institutionnelle et en perspective de carrière ça a été dit combien de remarquables à ESH de nos nos premières générations en quelque sorte, qui ont su construire un vrai savoir-faire un vrai savoir-et d'accompagnement ont dû se résout résoudre à abandonner pour trouver un vrai métier rémunérateur donc pour que les Oeuvres sache est un vrai métier, il leur faut un vrai salaire et un vrai service. Merci, cher collègue Madame Meunier. et qui sont dans une grande détresse celles et ceux qui ont assisté aux auditions que nous avons dû faire pour le projet de loi sur la CDU nisation a entendu leurs cris de détresse, on sait très bien ce qu'il viendra de ce que l'on peut voter dans cette assemblée, donc je me demandais si on ne trouvait pas le si on trouvait pas le courage pour dire, en les augmente, chacun prendra ses responsabilités après. Merci Madame Billon. Oui, et merci Monsieur le Président, moi j'ai entendu les arguments du rapporteur, j'ai entendu ce qu'a dit Monsieur le Ministre, j'entends bien entendu ce que dit notre collègue très engagée, Marie-Pierre Monnier, pour ma part je vais retirer cet amendement, je, je l'ai dit dans dans la discussion générale le budget est en augmentation, on part de très loin les AESH leur quantité et à la fois l'organisation progresse avec les pial même si il y a encore beaucoup de choses à faire à faire pour que l'égalité soit partout la même en terme d'application en termes de formation, donc, pour ma part, je retire cet amendement et j'espère qu'on va très très vite avancer sur ce sujet de l'accompagnement des 7 enfants en situation de handicap, je vous remercie. On ne 595 est retiré, je mets Madame Mellow. Monsieur le président je vais retirer aussi mon amendement qui est à peu près le même que celui de Madame Bio. Le 228 identique. Madame la présidente de l'aussi de 400 83 et retiré, donc je fais voter sur l'amendement 914 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté même vote pour 873 même vote il n'est pas adopté même vote pour 937 même vote il n'est pas adopté et donc nous passons à l'amendement 915 madame Dumas.

aux difficultés liées à la rémunération à la grande mobilité s'ajoute également une grande précarité de leur carrière le droit actuel prévoit que l'État employeur se doit de proposer un CDI au bout de six ans en CDD pour ces personnels, c'est trop long, ces personnels doivent être sécurisés, nous appelons à ce que les AESH soient recrutés en CDI, avec une formation adaptée dès le 1er contre, comme le proposait la PPL Victory examiné en début d'année à l'Assemblée nationale qui a été détricoté la stabilité de l'emploi est aussi un facteur d'attractivité, nous vous appelons à voter cet amendement qui débloque des moyens nécessaires à la titularisation des AESH. Collègue monsieur le rapporteur. La PPL devait l'être le l'occasion d'un débat approfondi et je suggère le retrait en hauteur dans la PPL. Merci, monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, vous proposer un plan de de titularisation massif des ASH à hauteur de 100 millions d'euros, je vous rejoins sur la nécessité d'assurer l'attractivité du métier des ESH c'est pourquoi, comme je l'ai indiqué nous les augmentons de de 10 pour 100, ce qui représente d'ailleurs une revalorisation de de 80 millions d'euros, qui est intégré pour 2023, j'ajoute que la création d'un corps de fonctionnaires auraient de nombreux inconvénients qu'il faut bien mesurer, y compris des inconvénients pour les AESH eux-mêmes, plus largement, une concertation, comme je l'ai indiqué y'lancer pour assurer aux AESH une à la fois une meilleure grille indiciaire et puis progresser vers les 35 heures, comme je l'ai indiqué

Jusqu'à récemment, l'état d'accompagnement des enfants en situation de handicap était pris sur le temps scolaire, périscolaire qui était à la charge de l'État, cette situation a été confirmée par plusieurs jurisprudences au motif Team que l'État le garant du service public de l'éducation et que ces temps périscolaire étant dans la continuité des heures de cours, ils relèvent donc du service public de l'éducation, cette situation cette situation au avait le mérite de la simplicité, or en novembre 2020, un arrêt du section du Conseil d'État est venue perturber cette situation en affirmant que désormais la responsabilité financière du temps fournis par les AESH devait être en prix, prise en charge par les collectivités, cette décision, en rupture avec l'idée et la pratique de ce qui se faisait jusqu'alors revient à un transfert de compétences de l'État, les collectivités sans compensation financière, or les collectivités n'ont pas toutes les moyens de prendre en charge ce temps fournis par les AESH au-delà de l'aspect juridique, monsieur le ministre, un enfant autiste qui doit être accompagné toute la journée, y compris durant le temps de la cantine scolaire et après les cours se bien de savoir si est dépendent de la collectivité ou de l'étape, son seul besoin, c'est d'être accompagné tout le temps et cela seul l'État peut peut assurer sans rupture d'égalité entre les situations et les territoires, nous étions donc avec cet amendement débloquer des fonds nécessaires à la réintégration des temps périscolaires dans le giron de l'État, si la question est de l'ordre législatif alors Monsieur le Ministre, proposez-nous une évolution de celle-ci, il nous serons ravis de l'étudier. Merci monsieur le président, dame de Marco, a rappelé le contexte mon amendement est profondément un amendement d'appel pour ne pas dire un amendement provocateur Les MDPH en effet indique très souvent que l'accompagnement de Neil sache doit se faire pendant le temps de la de la restauration scolaire pour que la scolarisation soit effective, sinon il n'y a pas de scolarisation, la commission des droits de l'autonomie des personnes en situation de handicap préconise également une prise en charge globale donc cet amendement monsieur ministre rappelle la nécessité d'assurer la continuité du temps de l'école qui, comme je le disais tout à l'heure ne se résume pas au temps temps de la classe si notre pays s'oriente enfin sur une politique de prise en charge de l'enfant, sur l'ensemble de la journée, on changera de logiciels on abordera la question se sous, sous une autre focale qui n'est plus celle de la scolarisation mais de l'accompagnement du handicap dans le temps de l'école qui est scolaire et périscolaire, alors Monsieur le Ministre, au travers de cet amendement, je souhaite tout simplement que l'on change de focale, la focale ne peut pas se réduire autant de l'école et ne peut pas non plus se réduire à par exemple, une proposition de CDI Sion des AESH pour penser voir régler la question, je crois qu'il faut une vraie politique globale continuer et partenariale de la prise de la en charge de l'enfant dans le temps de l'école, vous dites : concertation et conférence nationale mais j'avoue que pour l'instant, je vous vois peu peu en clair à changer réellement de focale, et c'est peut-être cela le sujet. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Le le président la la complexité du sujet qui, telle qu'elle apparaît au travers des amendements présentés avec beaucoup de conviction par Madame de Marco et par monsieur Brisson milite dans le sens de la commission des finances, qui est de demander le le retrait, en attendant que nous ayons une vision plus globale et que les collectivités locales s'exprime elles-mêmes, puisqu'elles ont très largement la responsabilité du temps périscolaire, qu'elle définit à la fois selon leurs moyens, et selon leurs propres politiques, nous avons donc des situations extrêmement différentes, c'est cette diversité que j'exprimais tout à l'heure pour formuler le voeu que si le sujet. Ne peut être que partagés et est rester un sujet d'actualité. et faisant le le la, un travail de préoccupation de tous nous ayons cependant le temps d'approfondir la complexité du sujet, je ne me sens pas capable de demander à l'Assemblée sur un amendement qui est un amendement d'appel pour monsieur Brisson, qui est un amendement plus construit sur le plan financier de Madame, de Marco pour traiter une question en en dessin. Passe de quelques minutes et en séance de nuit sur un sujet qui va impliquer la totalité des départements, par exemple, la totalité des des établissements donc je je souhaite le retrait ou sinon défavorable, non pas à raison de l'intérêt des sujets évoqués, mais en raison de l'incapacité de traiter ces sujets dans ces conditions. Merci monsieur le président, madame, monsieur, le les sénateurs, comme vous l'avez indiqué la responsabilité de la prise en charge pendant le temps périscolaire et en particulier pendant la pause méridienne des enfants en situation de handicap incombe aux collectivités, la décision du Conseil d'État et tout à fait clair à ce sujet, nous travaux dont nous travaillons donc dans dans ce cadre, à améliorer la la continuité des temps de prise en charge des élèves en situation de handicap, en particulier pour les élèves en situation autistique qui ont besoin d'une certaine continuité dans les dans les intervenants, mais l'ensemble sur l'ensemble des élèves en situation de handicap, seule une petite minorité, a besoin d'une continuité du temps scolaire et du temps périscolaire et donc cela se joue au niveau de chaque académie au cas par cas pour essayer de résoudre au mieux chaque situation, par ailleurs, le vote des crédits de crédit en en PLF n'aurait pas d'effet sur la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales déterminer par le législateur, par ailleurs, j'aimais donc un avis défavorable à ces amendements.

je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse simple à apporter à la question des AESH mais peut être comme ça en séquence en en scindant les difficultés en essayant de les traiter une par une, on améliorera la situation des ASH et on participera à cette professionnalisation de ce métier que je crois, nous, nous, nous souhaitons tous, en l'occurrence je j'ai entendu, expression, dire que c'est un amendement d'appel je je ne peux que l'inviter à à le retirer pour 2 raisons, et l'une qui comprendra très bien c'est que d'abord la commission culture, éducation et communication, a lancé une mission sur ce sujet et ça serait bien que nous attendions les résultats de du du travail que mènera notre collègue Cédric Vial avec l'ensemble de des membres qui voudront travailler avec lui, bien entendu, sur ce sujet et que nous soyons en mesure de faire des propositions concrètes au au Ministre sur cette problèmes d'articulation, pas si simple que ça, entre temps scolaire et périscolaire et puis deuxièmement, je crois que nous sommes tous conscients que ce n'est pas une décision budgétaire qui fera modifier la décision du Conseil d'État, on est sur un un un une une réponse qui est un autre ordre, me semble-t-il, à apporter, mais en tout cas merci pour vos amendements, ça permet d'aborder ce sujet, merci Monsieur monsieur le président, nous avons tous compris le sens de la décision du Conseil d'État qui est tout simplement à ce qu'est l'instruction obligatoire, le temps de l'instruction obligatoire, cela dit, le statu quo qui est né de cette décision du Conseil d'État n'est pas ne peut pas laisser en état de peut pas continuer aujourd'hui, il y a une grande diversité pour handicap identique entre un élève si qui est scolarisé dans une petite école d'une petite commune et un élève qui est scolarisé dans une école d'une grande ville, il y a une situation de de grande diversité entre d'établissement public, un établissement privé, on est aujourd'hui à handicap équivalent dans des situations de prise en charge de l'enfant qui sont caractérisés près du très grande diversité qui n'est pas acceptable au vu du handicap vous de l'avait cité tout à l'heure, quelques heures, monsieur le Ministre, donc il faut sortir de cette situation qui est une situation t'aime je pense que ça un mérite d'être discuté et cela mérite aussi d'ailleurs d'être discuté dans la Haute assemblée a coûté des travaux que vous ferez vous-même, il faut que le Sénat au delà de la de la mission flash de Cédric Jacques s'emparent de cette question de la prise en charge de l'enfant dans le temps de de l'école, donc je vous disais tout à l'heure monsieur le Ministre, qui a le temps de la classe, il y a aussi tout le temps de l'activité périscolaire, donc c'est une véritable politique de l'accompagnement de l'enfant en situation de handicap pour assurer ce que vous avez dit vous-même le continuum la continuité de cette prise en charge, je crois que les bonnes

si, il y avait un demande de retrait. Bon bé dans ces conditions, je vais retirer quand il est j'espère que ce sera remis au débat, quand même, c'est une préoccupation surtout des petites communes en grande difficulté. Si cher collègue, donc nous passons 875 Merci monsieur le président, en avril 22 le Conseil d'État a imposé le versement de la prime éducation prioritaire aux AUD exerçant dans les établissements concernés depuis le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que la prime serait également versée aux AESH, si nous nous réjouissons bien sûr de cette avancée pour ces personnels essentiels les projets des décrets à venir concernant les primes Rep et Rep plus pour les AUD et AESH ne prévoit pas les mêmes montants de prime que pour les autres personnels 3263 euros aurait et 1106 euros en REP, contre 5114 et 1734 euros pour les autres, rien ne justifie cette baisse des montants de prime pourtant fixe pour l'ensemble des autres personnels de l'Éducation nationale aussi, cet amendement vise à prévoir des crédits suffisants pour verser aux AESH et aux AUD, exerçant en établissement prioritaire, les mêmes montant de prime que ceux déjà versés aux autres personnels les auditions menées dans le cas des travaux préparatoires à l'examen de la proposition de loi des députés socialistes visant à lutter contre la précarité, des AESH et 10 AUD mise à jour les conditions extrêmement précaires d'exercices et de vie de ces personnels, les AESH perçoivent en moyenne une indemnité de 850 euros mensuels et vivent ainsi dans des conditions en dessous du seuil de pauvreté les à ED, quant à eux, avec l'équivalent d'un SMIC pour un temps plein qui n'effectuent généralement pas d'ailleurs, sont dans une situation à peu près comparables, ces personnels sont pourtant extrêmement investi, nous le savons dans leur mission est d'autant plus quand ils exercent dans les REP cet amendement pardon se propose ainsi d'augmenter de 11 millions d'euros, les crédits du titre de de l'action 03 inclusion scolaire des élèves en situation de handicap du programme 203 de l'élève, je vous remercie. Oui, monsieur le Président, la science de la commission des finances n'étant pas inépuisable et total, je demande l'avis du gouvernement. Merci, monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, madame la la sénatrice les jusqu'à présent, les AESH Elisa, ED ne bénéficier d'aucune prime en éducation prioritaire, nous créons cette prime, c'est une avancée significative en REP et 3711 euros brut annuels en re-plus ce sont des montants qui indique notre volonté d'améliorer la situation des AESH et des AUD, c'est un pas tout à fait significatif et dès lors j'émets un avis défavorable à votre amendement. Merci, Monsieur le Ministre, dont je mais aux voit cet amendement 875 avec 2 avis. Pour qui est pour, qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté 3 amendements discussion commune de 500 quatre Madame de Marco. Merci Monsieur le Président, cet amendement propose de renforcer les moyens alloués à l'enseignement professionnel, dont les crédits pour 2023 sont en baisse continue et l'inflation, les réformes successives n'ont cessé de réduire le nombre d'établissements, le nombre d'enseignants et le nombre d'enseignement, le projet de réforme du gouvernement sur les lycées professionnels semblent poursuivre une les mêmes actifs, l'enseignement professionnel est une voie d'excellence, si l'on donne aux établissements les moyens de fonctionner correctement, et si l'on valorise les métiers aux Californie. Merci monsieur le le le président je souhaite associer à cet amendement, ma collègue députée Fatiha Keloua Hachi puis le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, puisque comme vous le savez, ils n'ont pas pu n'ont pas eu la possibilité de discuter d'un budget aussi important que celui de de l'éducation en raison du du 49 3, donc oui concernant l'enseignement professionnel, vous savez que la réforme qui est en cours suscite beaucoup de craintes en raison de l'augmentation de la durée du stage au détriment de l'enseignement général et en 2021 2022, c'est ça un peu plus de 520000 élèves qui étaient accueillis en lycée professionnel, ce sont autant de de spécialités qui demandent un suivi spécifique et donc des moyens et un encadrement conséquent pour les lycées professionnels, or, non seulement les lycées professionnels ne bénéficient pas des mesures du gouvernement concernant l'apprentissage car les apprentis ne rentre pas dans leurs effectifs mais aussi en termes d'emplois les syndicats dénoncent des transferts de de la voie professionnelle vers la voie technologique et général, ainsi que des baisses horaires dans certaines disciplines, c'est pour ça que cet amendement propose d'augmenter les crédits ciblés sur les lycées professionnels de 25 millions d'euros.

alors Monsieur le Ministre, nous avons eu à l'initiative de nos collègues Les Républicains : débat sur l'enseignement professionnel, il y a quelques semaines de cela mais malheureusement au bout de 2 heures de débats, un certain nombre de nos questions n'avaient toujours pas trouvé réponse, et donc je me permets puisque l'enseignement professionnel est encore pour partie au moins sous votre responsabilité de vous poser à votre tour, ces questions rapidement, la première c'est comment fait-on lorsqu'on n'ajoute cinquante pour cent de à ce qui existe déjà dans l'enseignement professionnel pour maintenir un niveau d'enseignement théorique professionnel et généraux quand on sait que cet enseignement a déjà perdu 2 de nombreuses heures d'enseignement, de mémoire, je crois que en bac pro le français et l'histoire géo, c'est une heure 30 de cours par semaine, autre question lorsque les stagiaires vont aujourd'hui dans des entreprises, ils sont stagiaires et donc ils sont, ils ne perçoivent une gratification au titre de ce stage vos volontés voit le jour, ce seront alors des salariés dans les entreprises est-ce que vous pouvez nous éclairer aussi sur ce plan là, il nous semble que ça serait intéressant au moment où on parle de l'avenir de l'éducation nationale. Merci, cher collègue, monsieur le rapporteur. Monsieur le président de la commission des finances, a émis un avis défavorable, non pas que les les sujets soit inintéressant, mais comme le les intervenants l'ont précisé il y a une réforme de l'enseignement professionnel qui est préparé, nous attendons cette réforme pour en évaluer les modalités financières donc défavorable parce que prématurée, donc plutôt retrait sinon défavorable. Merci, monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, aujourd'hui près de 5 milliards d'euros sont consacrés à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et je rappelle que les professeurs de lycées professionnels sont également concernés par les hausses de de rémunération dont nous avons parlé précédemment, la réforme des lycées professionnels est en cours de d'élaboration avec des groupes de travail qui se réunissent depuis le 21 octobre sous la conduite l'égide de la ministre déléguée Carole Granjean,

en oeuvre et il sera concrétisé dans le futur projet de loi de finances 2024. En ce qui concerne les questions que vous soulevez, madame la sénatrice d'abord donc la réforme reste à écrire, nous avons réaffirmé d'une part le fait que les lycées professionnels bien dans les gîtes de l'éducation nationale, d'autre part, nous avons réaffirmé l'importance des savoirs fondamentaux dans la formation des lycéens professionnels, il n'y a pas de gratification actuellement pour les stages des lycéens professionnels, c'est quelque chose que nous envisageons pour l'instant ces gratifications n'existe pas et je vous rappelle également que la situation actuelle, c'est que, 2 ans après l'obtention du bac professionnel, près de la moitié des néo-bacheliers est au chômage, ça n'est pas une situation satisfaisante et c'est pour cela que nous nous attaquons à cette situation, des lycées professionnels, mais encore une fois la réforme est en cours pour toutes ces raisons, la réforme et puis. Les augmentations dont les professeurs de lycées professionnels bénéficient dans le cadre général du PLF 2023 j'émets un avis défavorable à ces amendements. Merci, monsieur le Ministre, donc je mais aux voix l'amendement 500 IV avec 2 avis défavorables. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté même vote pour ne s'en va même vote même vote pour 933 même vote, ils ne sont pas adoptés le 936 madame brûlant. Cet amendement vise à porter des crédits aux collectivités locales, qui ont à faire face à des dépenses énergétiques très importante pour les établissements scolaires communes pour les écoles, département et région pour les collèges et les lycées, c'est un peu du même ordre que ce qui avait été imaginé au moment du Covid ou parce que les protocoles sanitaires impliqués des dépenses supplémentaires pour les collectivités, l'État avait abondé de quelques crédits et nous en reprenons. Les mêmes sommes j'en profite Monsieur le Ministre pour vous interroger, très concrètement, voilà quelques heures que sont évoquées avec de plus en plus de de pression, je vais le dire comme ça, l'hypothèse la possibilité que j'espère, nous ne verrons pas mais que des coupures un délestage du réseau électrique soit opéré et que ça conduise à des coupures d'électricité, secteur par secteur, or dans ses chacun de ces secteurs, il y aura des écoles, des établissements scolaires, les préfets sont en train d'adresser des circulaires aux maires pour leur demander d'organiser les choses, il nous semble, je crois que vous rencontrez que votre ministère en compte les organisations syndicales enseignants demain à ce sujet, je crois que la représentation nationale, qui plus est, le Sénat, qui représente, entre autres, les élus locaux, a aujourd'hui besoin de savoir comment les choses sont envisagées toute la communauté éducative, les élus locaux ont très mal vécu les protocoles sanitaires qui était décidé le dimanche soir pour le lundi matin lorsque nous faisions face à l'épidémie à l'épidémie de Covid je crois que personne ne veut revivre ça, de même que nous ne souhaitons pas que les enfants et les jeunes qui ont eu de l'école par intermittence à cause de cette crise sanitaire et à nouveau de l'école par intermittence parce que leur établissement seraient les matinées visiblement privés d'électricité est-ce que vous pouvez nous éclairer, sans mauvais jeu c'est cher collègue sur la situation, Monsieur le Ministre. Merci, monsieur le rapporteur. ministère, le budget d'enseignement scolaire n'est pas le bon véhicule pour protéger contre la hausse du prix des combustibles et monsieur Ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice le la mission enseignement scolaire n'a effectivement pas vocation à porter ce type de dépenses en faveur des collectivités mais je rappellerai néanmoins que le gouvernement a mis en oeuvre une série de mesures à destination des collectivités locales, l'élargissement par amendement au PLF 2023 du filet de sécurité pour 1,5 milliards d'euros la DGF a également été augmentée de 320 millions d'euros dans le cadre du. Le PLF 2023 et puis 80 % des communes bénéficient du bouclier tarifaire, c'est-à-dire des tarifs réglementés de l'électricité, les collectivités qui ne sont pas concernés par le bouclier bénéficie de l'amortisseur tarifaire qui permet la prise en charge par l'État de 50 pour 100 des surcoûts, au delà d'un prix de référence, les collectivités bénéficieront aussi du fonds Vert, doté de 2 milliards d'euros, et enfin le président de la République a annoncé là un plan de rénovation des écoles qui permettra des rénovations notamment les chantiers dans le cas des rénovations thermiques sur la question, la 2ème partie de votre question, il pourrait, dans certaines circonstances, qui par nature ne sont pas prévisibles à l'heure actuelle, à savoir des périodes de froid très intense, le rythme de remise en charge des centrales nucléaires et les importations d'électricité, il pourrait en effet arriver que des délestages programmé comme la première ministre l'a indiqué puisse survenir en peau de léopard sur l'ensemble du pays ces délestages pourrait en effet concernés les établissements scolaires, mais les parents d'élèves et les élèves seront bien entendu prévenu de ces délestages qui pourrait intervenir le matin, selon 2 horaire 8 10 ou ou bien dix douze je mentionne également le périscolaire, le soir, qui est plus plus marginal de six heures à huit heures nous le faisons parce que sans électricité, les écoles et établissements scolaires ne peuvent pas accueillir les élèves dans des conditions de sécurité convenable, les systèmes de sécurité incendie seront ou seraient désactivés, il n'est pas possible d'accueillir des élèves avec des systèmes de sécurité incendie désactivé, c'est pour ça que, dans cette hypothèse-là et cette hypothèse est loin d'être je dirais envisager de manière certaine, au moment où nous parlons, il pourrait en effet être nécessaire d'organiser la rentrée des élèves en début d'après-midi, en incluant ou pas la pause méridienne et le repas à la cantine selon des une prévisibilité et une géographie que je ne peux pas déterminer à l'heure actuelle mais nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que les familles soient prévenues en temps et en heure. Monsieur le le ministre-je suis désolé mais je ne suis pas du tout rassuré par les explications que vous venez de donner d'abord bien sûr, personne d'entre nous ne souhaite ces coupures, on ne va pas se lancer dans un débat énergétique à à sept heures et sur cette mission Il y a un certain nombre de services régaliens, il y a un certain nombre d'établissements, je pense aux établissements hospitaliers qui vont être alimentés en permanence, pourquoi les écoles ne rentre-t-elle pas dans ce set. Là, pourquoi faut-il imaginer que nos élèves vont devoir rater des cours parce que l'électricité va manquer ensuite vous dites les parents seront prévenus d'après les informations que j'ai, ils vont être prévenu la veille pour le lendemain et on va se retrouver avec des parents qui vont amener leurs enfants devant les écoles et des mères qui vont être obligés de se débrouiller de la situation et je pense qu'il faudrait travailler très sérieusement sur cette situation et ne pas aller dans les pistes que vous évoquez, parce qu'on va au devant de très graves problèmes me semble-t-il. Merci, cher collègue, donc je mais aux voix l'amendement 936 avec 2 avis défavorables. Qui est pour, qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté 2 amendements discussion commune 883 Madame Monnier. Merci, donc cet amendement vise à revenir sur la baisse des 1117 TP dans le 1er degré public pour la rentrée 23 à rebours de la priorité primaire au primaire mise en avant par le gouvernement depuis 2017 cette suppression apparaît difficilement compatible avec la poursuite des politiques de dédoublement en rai près plus CP-CE1 grande section et le plafonnement à 24 élèves à 24 élèves par classe, si les objectifs affichés de ces politiques sont louables, ces dernières ont un coût en ETP important qui a été lors du précédent quinquennat absorber en partie par le redéploiement des ETP précédemment mobilisés dans le dispositif plus de maîtres que de classes et mais aujourd'hui il est exsangue, le ministère justifie cette suppression par la baisse des effectifs cet argument rencontrent pourtant ses limites quand on sait que la France a fait encore par fait encore partie des pays européens avec le plus d'enfants par classe en primaire, 19 élèves contre 13 virgule cinq en moyenne dans l'UE 15 en Allemagne 12 en Belgique, en Italie, cette baisse de poste risque par ailleurs de conduire à des fermetures de classes, lourde de conséquences pour nos territoires ruraux, ainsi qu'un non-remplacement des personnels absents pénalisant, aussi bien les classes que les formations continues sur le temps de travail. C'est également un amendement qui vise à empêcher la suppression des 1117 postes dont la suppression est prévu dans le 1er degré public aux arguments qui viennent d'être développés par Marie-Pierre Monier je voudrais effectivement ajouté que les objectifs de dédoublement, grande section, CP, CE1. En rai plus devait être atteint au quinquennat précédent, de même que les 24 élèves pour toutes les autres classes et dans les secteurs or REP, ça n'est pas le cas, à ma connaissance, il y a près de 90000 classes encore où les effectifs sont supérieurs à 25 élèves, ce qui reste très important, et puis on l'a tous régulièrement souligné ici, il y a un sujet de remplacement et un nombre très conséquent d'enseignants qui sont absents pour maladie, formation etc. Ne sont pas remplacés, il serait d'ailleurs intéressant de calculer combien cela représente d'heures de semaines de mois de cours dont les élèves sont privés et je crois que dans le Grenelle organisé par votre prédécesseur, monsieur le Ministre, il a été question à juste titre de renforcer la formation continue des enseignants, ce qui est très juste, mais alors il faut développer les moyens de remplaçants bon sinon à chaque fois qu'un professeur ira se former, ce sera une classe qui se trouvera privé d'enseignants. La commission des finances est défavorable et je partage son sentiment de c'était les effectifs doivent évoluer avec les effectifs les enseignants, avec les élèves. Monsieur le président, les madame la sénatrice les suppressions prévues prennent acte de la baisse des effectifs scolaires, en particulier dans le 1er degré le dédoublement des CP et ses vingt et tu achevé aujourd'hui, il nous reste à poursuivre le dédoublement des grandes sections de maternelle qui être achevé, auteur de 74 le taux d'encadrement dans le 1er degré va s'améliorer puisque nous allons passer de 21 virgule 6 à 21,3, par conséquent je ne retient pas votre amendement.

Oui. Cet amendement, il vise à apporter, en fait, des moyens supplémentaires au personnel d'éducation CPE à ED surveillant d'externat, sont autant de fonctions essentielles au bon déroulement de la scolarité d'un élève pourtant depuis 2017 on compte au total 1914 personnes d'éducation en moins, ce sont 1300 à ED en moins 400 CPE en moins, le recrutement de 100 CPE pour 2023 ne suffira pas à combler la perte sous le quinquennat de François Hollande, ces personnels avait pourtant vu leurs effectifs croître de 2518 café le gouvernement sous le précédent quinquennat pour perte c'est personnels si essentiel à la vie scolaire, cet amendement vise à revenir aux effectifs de 2017, conscient que l'enjeu reste le manque d'attractivité pour ces métiers, c'est pour ça que nous demandons une revalorisation des salaires de ses personnels d'éducation. Avec les bons sentiments ne font pas la bonne politique budgétaire et que les résultats de la gestion du quinquennat de Monsieur Hollande ne prouve pas que cette augmentation est régler les problèmes de notre école. Donc c'est défavorable. Monsieur le Ministre. de mesures de revalorisation et par ailleurs les à ED, comme vous le savez, bénéficieront des primes rep plus ce qui n'était pas le cas par le passé et j'ajoute que depuis la rentrée 2019 les AMD qui préparent les concours pour devenir enseignant, peuvent bénéficier d'un contrat de pré-professionnalisation pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable. Je mais voit le 800 90 avec 2 avis défavorables. Qui est qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté de 911 monsieur prennent. Oui, la formation des enseignants comme vous le savez, doit être de qualité dès l'entrée dans la profession, mais aussi tout au long de la carrière pour permettre un approfondissement sérieux des contenus didactiques et répondent à des besoins ciblés par les équipes selon leur problématique et leur aspiration personnelle, cela est un besoin identifié au sein de la profession 76 % des enseignants déclarent effectuer des tâches pour lesquelles ils auraient besoin de plus de formation et cela conditionne bien évident, la réussite de tous les élèves, ce besoin de moyens pour la formation continue et d'autant plus important que la réforme de la formation initiale, instaurée par le gouvernement sous le précédent quinquennat consiste à confier une classe à un enseignant stagiaire sans accompagnement, une technique de pré-titularisation qui permet au ministère de justifier la suppression de postes d'enseignants afin de répondre à la crise des vocations, il est nécessaire de développer une politique de formation continue ambitieuse en 2020 la loi de finances diminuer ses crédits de près de 30 millions d'euros, il est donc proposé tout simplement de rétablir ce montant pour répondre aux besoins. je dis bien et là ces crédits de formation permanente ne sont pas utilisés dans la totalité des lignes ouvert, ce qui prouve que le problème de la formation des enseignants n'est pas fondamentalement un problème financier mais un problème d'organisation et d'orientation. Merci, monsieur le Ministre. une augmentation de 100 millions d'euros par rapport au budget 2022 c'est une enveloppe ambitieuse qui permettra de financer une formation continue sur laquelle, par ailleurs, nous réfléchissons quant à son contenu, il y a son organisation dans ces conditions j'émets un avis défavorable à votre proposition. des sujets de divergence que nous avons avec vous et qui explique l'abstention que nous souhaitons de certains nombres dans nos rangs, ce qui pas vous vous vous augmenter le budget et puis vous dites nous allons réfléchir à une autre organisation, est ce qu'il aurait pas été souhaitable que la réflexion sur l'organisation, soit se fasse en même temps que l'augmentation du budget curieuses pratiques de politique que d'augmenter des moyens de mettre toujours plus de moyens et de réfléchir après c'est peut-être cet été, jamais à l'organisation du site.

Cet amendement vise à renforcer les moyens des Rased, de la maternelle et de l'école à la élémentaires, les professeurs spécialisés, les psychologues scolaires sont des renforts très importants aux équipes enseignantes et aux parents malheureusement les alertes se multiplient dans un certain nombre de territoires sur le manque d'effectifs, de ses réseaux en forte dégradation depuis plusieurs années, le nombre de Rased n'a pas augmenté a même légèrement diminué depuis 10 ans, nous souhaiterions donc un moratoire s'appliquant à la fermeture des postes en Rased soient appliquées, ainsi qu'une carte des renforts nécessaires en lien avec le collectif national des Rased, cet amendement tend donc à octroyer 30 millions supplémentaires au développement de ces Rased. Monsieur le rapporteur. Commission demande le le retrait, considérant qu'il n'y avait pas une nécessité absolue. Merci, monsieur le Ministre. Monsieur le président, madame la la sénatrice les moyens mis en oeuvre au travers des Rased, qui représente 10300 emplois pour 2021 2022, ce sont des moyens stables qui répondent aux besoins, par ailleurs, nous poursuivons le dédoublement des classes en éducation prioritaire du côté des grandes sections des écoles maternelles ou encore pour la mise en oeuvre de l'instruction de l'éducation obligatoire à partir de l'âge de 3 ans, compte tenu de ces éléments un abondement budgétaire supplémentaire n'est pas nécessaire : avis défavorable. Merci donc je mais aux voix l'amendement 877 avec 2 avis défavorables. Qui est pour, qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté 3 amendements en discussion commune de 879 madame nègre. Oui, monsieur le président, cet amendement vise à revaloriser les métiers de la médecine scolaire, alors que la France ne compte déjà qu'un médecin pour 12572 élèves et un infirmier pour 1300 élèves, les effectifs de ces personnels de santé, de l'éducation nationale sont en chute libre depuis 2017 on compte moins 30 % de médecins et moins, moins 11 % d'infirmiers dans le milieu scolaire, la raison de nous la connaissons toutes et tous, le manque d'attractivité de ces métiers liés à la faible rémunération et à la prise en charge de plusieurs établissements pourtant le besoin de médecins, d'infirmiers, de psychologues est cruciale dans le milieu scolaire pour a suivi pour assurer le suivi médical des élèves et le repérage des situations relevant de la protection de l'enfance, le service de la médecine scolaire fonctionne si mal que nous sommes ici nombreux à vouloir la confier aux départements, cet amendement propose donc une revalorisation salariale des métiers de la médecine scolaire, afin afin de rendre plus attractifs ces métiers et ainsi donner secteur les moyens de lutter contre les inégalités sociales de santé au sein de l'école et nous proposons donc une mesure de 30 millions pour la revalorisation de ces personnels. Oui, merci Monsieur le Président, la situation de la médecine scolaire est de plus en plus critique à l'image des chiffres présentés dans ce projet de loi de finances 2023 il y avait 1271 médecins scolaires en 2012, il n'y en a plus que 843 et dans 19 départements, il y aurait plus de 20000 élèves sur la responsabilité d'un seul médecin donc, vous l'avez compris, ça a été déjà dit il y a une urgence, elle n'est pas nouvelle Monsieur le Ministre, bien entendu, il faut trouver des solutions le le salaire ne sera pas la seule solution pour rendre attractif le métier, nous sommes tous issus de territoires où les déserts médicaux nous occupe à plein temps, si je puis mince primaire ainsi je, je, j'appuie cette urgence sur la médecine scolaire, parce que, et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons rendu notre rapport porno l'enfer du décor qui dresse un tableau extrêmement grave sur l'industrie de la pornographie, mais aussi sur l'accès des mineurs et sur l'éducation à la sexualité cette médecine scolaire peut contribuer aussi à prévenir à faire du suivi médical et à recevoir la parole de ses enfants, il est question, peut être aussi, on peut évoquer aussi la prostitution des mineurs, puisque, à 10000 mineurs se prostituent aujourd'hui en France, il faut les repérer pour pouvoir les accompagner et la médecine scolaire, bien entendu, un rôle à jouer, je vous remercie. les médecins scolaires, pour rendre cette profession attractive et combler les manques que nous connaissons aujourd'hui et en complément de ce que viennent de dire nos collègues, je voudrais insister sur les nombreuses études qui montrent qu'après la période de crise sanitaire que nous venons de vivre les enfants et les jeunes sont dans une santé mentale et psychique dégradé et qu'il y a besoin plus que jamais de renforcer la médecine et la santé scolaire. Merci, monsieur le rapporteur. Commission des finances, a donné un avis défavorable que je vous rapporte avec conviction parce que je pense très honnêtement que la démographie médicale est un problème général, on ne trouve pas non plus de de médecin du travail, par exemple, nous ne le règlerons pas par ces amendements sur des sommes qui sont à la fois importante pour le budget est insuffisante pour modifier ces questions de démographie médicale qui paralyse tout et qui préoccupe tout le pays, je vais faire du Brisson dans le texte, on va réfléchir avant de dépenser. Merci, monsieur le Ministre. Monsieur le président, je partage le point de vue du rapporteur, j'ajoute que qu'une qu'un travail est actuellement en cours, menée par 3 inspections générales Lygia l'IGAS et l'IG ESR qui devrait nous offrir une perspective sur la situation de la médecine scolaire, car nous avons revalorisé de manière significative les médecins scolaires, avec une augmentation de 45 % des de et de fonctions et d'expertise en en 2021 et 2022 nouvelles marges de revalorisation des médecins est prévue au PLF 2023 c'est vrai également du côté des infirmiers le la, le, le, on a un et un rendement des concours qui est satisfaisant du côté des des infirmiers avec des campagnes de communication qui ont été menées du côté des écoles d'infirmiers et d'infirmières et quant aux psychologues scolaires, leur nombre a augmenté de plus de 7 % entre 2017 et 2021, nous prévoyons une enveloppe assez substantiel revalorisation de 6 8 millions d'euros pour 2023 pour les médecins, les infirmiers et les psychologues de l'Éducation nationale pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable à cet amendement. Et je mets aux voix le l'amendement 879 de Madame Monier avec 2 avis défavorable qui est pour.

je le retire parce qu'il n'a pas tellement de chance d'être adoptée, en réalité, il y a, il y a, il y a eu des alertes depuis de nombreuses années, il y a la situation dans les territoires avec ce déficit de médecins, on est bien entendu convaincus que vous n'allez pas trouver des médecins comme ça du jour au lendemain, vous n'avez pas de baguette magique, nous non plus, donc ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est que dans les territoires, aujourd'hui il y a cette situation de déficit de médecins mais il y a des solutions innovantes qui sont aussi mises en place pour pouvoir pallier donc il besoin de trouver des solutions, des solutions innovantes pour mettre à disposition, peut être par exemple dans les déserts médicaux, il y a désormais des sages-femmes qui s'installe dans de toutes petites communes et qui pallie au déficit de gynécologues médicaux dans les territoires, donc moi j'aimerais qu'on puisse apporter déjà des solutions innovantes pour essayer de d'amortir cette situation qui est quand même dramatique pour les enfants, je vous remercie. Qui s'abstient, il n'est pas adopté 2 amendements discussion commune 935 monsieur Julia. Merci monsieur le président, monsieur Miss mais mes chers collègues, cet amendement porte sur les effectifs du du second degré

rapporteur pour la commission de de la culture, ça lui permettra peut-être de de s'exprimer maintenant qui disait très très justement dans son rapport que l'an passé, il y avait eu 12 millions d'euros d'heures supplémentaires non consommés, donc votre ministère, Monsieur le Ministre, met en place une politique d'heures supplémentaires pour compenser le manque de postes, mais manifestement elle ne fonctionne pas parce que les professeurs ne souhaite pas obtenir ces heures supplémentaires, donc il faut changer les les façons de faire et la solution, c'est sans doute de rajouter des effectifs, merci monsieur le président. Oui, cet amendement vise à rétablir les 481 ETP supprimés dans l'enseignement secondaire pour ce PLF 2023, il faut rappeler que 7500 emplois ont été supprimés dans le secondaire entre-2018 et 2021, malgré une hausse des effectifs de 68000 élèves la baisse de 5000 élèves que l'on enregistrera en 2023 ne justifie donc pas de supprimer encore des postes, elle constitue seulement un espoir de voir les conditions de travail des élèves et des enseignants s'améliorer légèrement car les conséquences des suppressions de postes de ces dernières années se mesure sur le terrain dans le département de la Drôme, par exemple, elles sont très concrètes, ces établissements ont connu une ou plusieurs fermetures de classes difficiles, ce qui signifie des effectifs élevés et donc de moins bonnes conditions de travail pour élèves et enseignants des postes supprimés, cela signifie aussi moins d'adultes présents dans l'établissement et donc moins d'accompagnement et de projet pour les élèves, l'expérience nous montre que nous manquons déjà de poste, vous propose de renoncer à en supprimer davantage. Défavorable, c'est contraire à la politique de la commission des finances, qui souhaite que les effectifs soient atteints à 2 adapté pardon aux besoins en élèves du secondaire. Si Monsieur Ministre. Monsieur le président, madame la sénatrice le le budget prend en compte la baisse de 10400 élèves dans dans le second degré et le schéma d'emplois proposées en PLF 2023 garantit la stabilité du taux d'encadrement dans le second degré et pour ces raisons, j'ai mis un affût un avis défavorable. Merci donc je laisse aux voix l'amendement 235 avec 2 avis défavorables. Qui est pour,

Merci monsieur le président, messieurs le ministre monsieur le rapporteur, cet amendement et les 14 suivant concerne donc l'installation de jeunes agriculteurs formé et dans l'enseignement agricole 900 82, la France comptait 1 virgule 6 millions d'exploitations agricoles, il y en a aujourd'hui 416000 en 40 ans, la France a perdu donc 30000 exploitations par an, c'est-à-dire une exploitation par an et par commune, si je me rapproche de l'Aveyron, mon département, il y a encore cent quarante ans 100 80 jeunes qui s'installe à l'agriculture, mais il y en a 300 qui arrête et même si nous partagerons être de département caisse talent le plus avec quelques départements bretons et les Pyrénées-Atlantiques : c'est quand même dramatique dans le renouvellement des générations, et donc d'enjeu stratégique pour la France pour sa souveraineté alimentaire pour le maintien de nos paysages ouverts, on va le dire comme ça, pour une France des terroirs vivante pour une France rurale comme nous et bon et donc pourrait 20000 agriculteurs par an contre 13000 aujourd'hui, il est indispensable, donner les moyens à l'enseignement agricole et donc mon amendement comme les autres vise finalement est un amendement d'appel, pas d'appel au secours, mes appels pour veiller à ce que effectivement l'enseignement agricole et les moyens de pouvoir former ces jeunes qui seront la France de demain. Défendu le 600 Madame bidon. Merci monsieur le Président, évidemment, les amendements ont été défendu l'idée, c'est forcément de donner plus de moyens à l'enseignement agricole, on le sait, c'est un enseignement performant, pas suffisamment connu d'ailleurs et a suffisamment connu de dans l'orientation pour les les enfants et les familles, donc : donner plus de moyens, l'agriculture en a besoin de nombreux la moitié des agriculteurs vont partir dans les années à venir à la retraite, il faut les remplacer, il faut des compétences donc donnons-nous les moyens de former ses compétences, je vous remercie. Merci, 2 amendements identiques : le 876 madame Meunier, défendu le 941 monsieur Nick. Oui, donc, cet amendement de mon collègue Joël Labbé vise lui aussi à soutenir l'enseignement agricoles à hauteur de 29 millions 200 25, donc ça a été dit, outil essentiel pour notre agriculture nos territoires, on a besoin de former les agriculteurs avec le renouvellement des générations 250000 exploitants arriveront à l'âge de la retraite en 2000 26 et nous installons aujourd'hui seulement 13000 nouveaux agriculteurs par an, c'est aussi un enseignement public fort pour assurer la transition agroécologique essentiel là. là. 142 c'est un amendement de repli. Deux est un amendement de repli par rapport à celui-ci, qui vise à rétablir la situation, à hauteur de 15 millions 200 52 pour revenir sur les suppressions de postes massives de ces dernières années. Merci de 880 Madame Monier défendu. J'ai fait. Défendu le 235 Monsieur Anglade. L'amendement 245 dans le même objectif simplement de donner les moyens de TP pour réaliser l'objectif que j'ai indiqués pour la formation des jeunes. Merci de 881 madame Monnier. la récente réforme du lycée, repose en partie sur la variété des enseignements pour être choisis par les élèves dans l'enseignement agricole public la baisse continue des ETP, mais aussi des dotations depuis plusieurs années, ne permet pas d'assurer l'offre minimale de 30000 heures d'enseignement facultatif L'inea le minimum d'une option par lycée mentionnés par les référentiels programme y compris pour les matières les plus essentiels dans cette formation, comme les mathématiques ou l'agronomie, donc l'enjeu c'est de rétablir 4 ETP, cet amendement pour préparer les élèves de l'enseignement agricole public à la transformation de nos systèmes agricoles et alimentaires, leur offrant des possibilités variées de développer leurs connaissances et leur savoir-faire mais aussi plus simplement d'assurer dans chaque lycée, les enseignements de base nécessaires à la préparation du Baccalauréat.

Est ce que beaucoup de salariés accepteraient de travailler une heure payer une demi-heure, hé bien non, et c'est pourtant ce qui se passe. Pour l'accompagnement personnalisé pour les élèves de la filière technologique agricole, donc il est proposé par le présent amendement le rétablissement de ces vins et qu'il avait en équivalent temps plein pour la rentrée 22 23 pour établir de façon pérenne le paiement d'une heure, payer pour une heure fait je crois qu'il y avait eu un engagement de la directrice générale de l'enseignement une réponse du gouvernement, paru au JO du 1er septembre 2020 ou il est reconnu, qu'il s'agit bien ici d'heures d'enseignement et nombre d'heures supplémentaires occasionnel depuis l'engagement n'a pas été confirmée dans les faits,

Oui, merci Monsieur le Président, donc il est toujours question de de moyens humains pour l'enseignement agricole et notamment de TP à destination d'une matière importante, c'est enseigner, promouvoir les valeurs de la République, notamment les valeurs civiques et en fait dans les classes de seconde professionnelle des lycées agricoles publics ces ces heures ne ne figure pas, n'existe pas, donc c'est pour combler cette lacune, je vous remercie. Merci le 939 Madame brûlant ou monsieur aux US. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, oui c'est une une grosse lacune dans l'enseignement agricole, aujourd'hui il n'y a pas de d'enseignement sur les valeurs de la République, on avait eu des débats très fort ici et chers collègues, vous, vous vous y avez beaucoup tenu et ce qui manque surtout, c'est des des horaires dédiées à à tout ce qui concerne l'instruction civique, alors en 2022 Monsieur le Ministre, faute de moyens, vous avez essayer de grappiller sur différentes disciplines pour mettre en place de façon très précaire cet enseignement, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est des postes de titulaires pour pouvoir l'assurer réellement ça serait complètement incompréhensible que dans les lycées agricoles, il puisse pas y avoir une une instruction civique comme dans les autres classes, merci monsieur le président bonjour. Merci le 882 madame Meunier. Donc, cet amendement vise à rétablir ne partir des emplois supprimés depuis 2019 dans l'enseignement technique agricole qui permettaient d'assurer les dédoublements obligatoire dans les établissements, le Conseil général alimentation de l'agriculture des espaces ruraux reconnaissait dans un rapport remis en vain que la réforme des seuils des doublement dans l'enseignement technique agricole était avant tout lié à la diminution du nombre de TP dans les établissements et décidé en parallèle par le gouvernement, ainsi les seuils de dédoublement des classes, en plus d'être augmenté 3 élèves sont devenus indique. Et non obligatoire, est de retour, qu'on a sur le terrain, ça met parfois en danger les élèves particulièrement quand ils sont. à deux travailler avec les grands animaux n'avait tant dis donc l'autre objectif annoncé de cette réforme était de soutenir l'augmentation des effectifs d'élèves de l'enseignement technique agricole, leur seul moyen d'Athènes dans cette cible est au contraire d'assurer le maintien d'effectifs et de moyens pédagogiques l'enseignement des groupes réduits, quitte à ouvrir une nouvelle classe dans les établissements permet après de tissage de qualité mais aussi un meilleur respect de conditions de sites, sécurité, en particulier dans les lors des travaux dirigés. Merci, monsieur le rapporteur. Sur ces 14 amendements. Ben oui, il y a 14 amendements et qui ne sont pas tout à fait identique, mais la commission des finances à bord, on a une immense, une grande sympathie pour l'enseignement agricole, monsieur le ministre de l'Agriculture, le l'enseignement agricole quadrillent nos territoires, qu'il s'agisse de l'enseignement public des lycées agricoles, qu'il s'agisse de l'enseignement privé et notamment des maisons familiales rurales, nous sommes très attentifs, on on a, il y a d'ailleurs un effort significatif qui a été fait cette année. Et qui malheureusement ne s'accompagne pas d'une augmentation identique à proportion des élèves et en toute la question, c'est la poule et l'oeuf, on commence par quoi est-ce qu'on est, on a une offre d'enseignement qui d'ailleurs n'est pas simplement agricole mais qui est rural et surtout les métiers de la ruralité dans l'immense majorité des cas. Sentiment un préjugé favorable et-ce une nécessité absolue, je demande l'avis du ministre. Merci, monsieur le Ministre. Les amendements globaux, après on pourra entrer dans le l'enseignement civique et la communication. D'accord. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, monsieur le rapporteur spécial, madame, monsieur le rapporteur pour avis dans messieurs les sénateurs, Monsieur le Ministre, je suis, je suis très heureux d'être ici ce soir pour évoquer la question l'enseignement agricole ça prouve, et c'est ce qu'on voulait démontrer aussi avec mon collègue PAP Ndaye d'abord le la reconnaissance de la diversité et la spécificité de l'enseignement, école et au fond, la volonté que nous avons tous les deux et le gouvernement tout entier, de faire en sorte que chaque jeune puisse trouver sa voie, alors je j'essaye de répondre à l'interpellation du rapporteur spécial longuet sur un certain nombre de sujets, je ne sais pas si vous voulez que je fasse tous les ans on on peut être de dire la question des effectifs, une somme, c'est pas la c'est pas forcément la question de la poule et l'oeuf, alors on a eu un une une légère diminution des effectifs scolaires, on a une légère augmentation des effectifs en apprentissage, ce qui fait que globalement on a plutôt des effectifs qui sont en augmentation, on est logé à augmentation des effectifs ou une stabilisation des effectifs d'enseignement et pour répondre à la question du de votre rapporteur, l'objectif est bien de faire en sorte qu'on mette en adéquation les besoins des élèves et les effectifs qu'il faut mettre en face c'est c'est bien ça que nous essayons de marquer cette année, je voudrais juste rappeler, Monsieur le Président, quand même, que l'enseignement agricole, c'est d'abord les 18000 agents du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, les plus de 800 établissements, ça a été dit par l'Europe, votre rapporteur qui sont très présents dans les territoires, c'est un ancrage territorial qui est très précieux, me semble-t-il, les 155000 élèves scolaire 7000 apprentis, les seize mille qui sont en enseignement supérieur, c'est-à-dire la variété, la diversité des métiers et les 200 métiers qui sont exercés qui sont enseignées pardon dans ces établissements, c'est donc la variété de ses enseignements avec un taux de réussite qui est très exceptionnel que beaucoup salué et dont je voudrais aussi au travers de cela saluer la qualité de l'enseignement et au travers de ce budget, nous avons essayé plutôt d'encourager les équipes pédagogiques qui sont très mobilisés dans une logique souvent très inclusive dans ses établissements scolaires peut être que je commence par les amendements identiques sur la question des moyens 234 600 à 876 941 il me semble que pour toutes ces raisons, faisant écho aussi à ce qu'a dit le sénateur Brisson, on met des moyens à la hauteur de ce que sont les besoins des élèves, on aura des éléments, ça a été dit par un certain nombre d'entre vous, donc, au travers de la loi d'orientation agricole, il me semble que là, permettez-moi cette expression qui qui comme un gant à l'enseignement et quand il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs, il me semble que la question n'est pas tant d'abord de se poser la question des effectifs et de la l'attractivité c'est l'attractivité du métier qu'il faut d'abord travailler, c'est la question de la rémunération, ce qu'on a évoqué hier soir, ne lever un certain nombre de contraintes et de faire en sorte que le métier soit attractif dire aussi, me semble-t-il, me semble-t-il pour la la sénatrice Billon que les éléments de communication font quand même que c'est un enseignement qui est plutôt attractifs dans une démographie que vous avez évoqué en début des échanges, avec mon collègue PAP Ndaye qui qui est décroissante, on a des effectifs qui sont en croissance, même légère, d'un peu plus de 1 % et donc on a quand même quelque chose qui attractifs, donc les stratégies de communication me paraît aller dans la bonne direction et c'est dans la loi, effectivement, d'orientation et d'avenir que nous traiterons aussi la question de regarder globalement ce que sont là les les moyens de faciliter l'arrivée de et l'attractivité des métiers et le fait que un certain nombre de jeunes s'orientent vers ces métiers, je dis au passage Madame d'abord c'est un enseignement qui est quasiment paritaire, il y a plus de jeunes femmes que de jeunes hommes qui sont dans cet enseignement et pour vous donner un élément complémentaire d'appréciation c'est moins 4 pour 100 de tête sur les métiers de service pour les jeunes femmes et plus 5 % pour les jeunes femmes sur les métiers de production, c'est dire que la tendance que vous souhaitez étant va plutôt dans le bon sens, enfin je dis un mot du budget puisqu'on est sur le budget, c'est les moyens en effectifs des personnels, c'est aussi les moyens en ressources humaines, je suis, je suis sûr qu'il ne vous a pas échappé qu'on a, on a une 36 emplois qui sont créés sur le programme de 215 et dans ces 36 emplois des effectifs qui vont être affectés environ au service des ressources humaines, parce que quand j'ai rencontré les organisations syndicales, avec mon collègue Pap Ndiaye on essaie aussi de regarder, d'écouter, d'ajuster les dispositifs, on a bien vu qu'il avait un sujet de ressources humaines, au-delà du cas particulier qui n'est pas normal, on a bien une sujet de tension, il faut faire grief à personne, sauf qu'il faut qu'on essaye de répondre aux questions et aux sollicitations et donc sur ce sujet-là, voilà ce que nous allons faire et donc c'est bien intégrer dans les moyens et les Budgets, ceci étant dit, sur l'ensemble des éléments, il me semble que le budget est bien ajusté, donc c'est une demande de retrait pour les amendements que je viens de citer, sinon c'est un avis défavorable. Et sur les autres.

Le 876941. D'accord, et de 942 aussi oui. Et du coup, monsieur le rapporteur, qui avait demandé l'avis du gouvernement, a le même avis. Oui, moi je, je crains malheureusement qu'au nom de la commission des finances je ne puisque demander le retrait de ces amendements. tout en formulant le voeu que les besoins soient satisfaits, ce qui, mais parce que c'est vraiment un enseignement qui quadrillent notre territoire et dont la polyvalence, c'est un vrai succès, je ne voudrais pas que des des élus territoriaux ne disent mais vous nous avez privé de moyens dont on avait besoin, or manifestement, ce n'est pas le cas à cet instant. Dans ce cas-là, je je demande aux auteurs des amendements d'augmentation à 29 millions 15 millions et 3 millions de retirer en sachant que nous avons en quelque sorte un otage le ministre. Sur l'agriculture qui est venu pour la première fois défende sa mission et qui nous dit : avec les 70 millions de plus de cette année, je boucle mon système et je dis non à personne.

parce que il y a 14 amendements en discussion commune c'est donc c'est sur tous les amendements monsieur voilà. Monsieur le Ministre du coup sur les autres amendements. Pardon, monsieur le président, monsieur le rapporteur, alors du coup je réponds sur les autres amendements confirmant ce que j'ai dit sur le fait que nous ajustons les moyens au mieux de ce qui nous paraît être les besoins, les besoins du territoire il y a une stabilisation, voire une légère augmentation des effectifs, il me semble important

du travail qu'elle a fait en commission, je vous cherchez madame la sénatrice si vous bougez de place évidemment à cette heure-ci, ça va me compliquer la tâche, vous remercie du travail que vous avez fait en commission et saluer ce que vous avez dit sur un certain nombre de points à la fois de vigilance et de point budgétaire et je crois qu'on a eu un échange je dis soleil du de votre président de commission qui a été fructueux et qui a permis d'éclairer un certain nombre de sujets qui a permis de montrer, je crois que nous avons et ça répond à la question de votre rapporteur spécial des moyens qui sont bien engagés, donc sur les 450 retrait sinon défavorable sur les autres employes sur la question des moyens, les emplois supprimés, le rétablissement des emplois supprimés reconnaissance ça été dit d'ailleurs par vos rapporteur successivement, phase de diminution des effectifs à l'époque en net, c'est moins que ce que vous et que vous annoncez, mais il me semble que là on est dans un autre moment de stabilisation stabilise les effectifs et là où il y a une forme de cohérence et donc c'est un avis demande de retrait sinon un avis défavorable sur les questions qui a été posée par la sénatrice Monnier sur la question de rétablissement des effectifs, il me semble que, comme on l'a vu dans les amendements précédents relatifs aux humain, je vous confirme que les suppressions était corrélée à la diminution des effectifs et on je vous assure que les référentiels et les volumes horaires prévus dans l'accompagnement personnalité sont respectés, que les élèves de la voie technologique en bénéfi tous bénéficient tous et 878 demande de retrait sinon défavorable, madame la sénatrice Billon sur le soutien à la l'enseignement moral et civique juste vous rappeler que c'est en fond Edgar Pisani, c'était un certain temps mais c'est souvent d'actualité, Edgar Pisani, surtout quand on est ministre de l'Agriculture, c'est quand même une figure du ministère de l'Agriculture au couche souvent à qui beaucoup de monde se réfère

d'échanges internationaux, donc ils ne sont que les crédits qui sont déployés les stratégies qui sont déployés, souvent en autonomie d'ailleurs assez grande des établissements sont suffisantes et donc il y a pas besoin de rajouter des crédits, donc sur ces deux amendements 600 et 900 39 retrait sinon défavorable, enfin, sur le dernier amendement de Madame Mounier c'est un du monde de retrait, sinon c'est un avis défavorable. Merci madame brûlant. Vous vouliez intervenir non non. La présidente. Le. Oui, merci, je n'avais pas défendu tout à l'heure, l'amendement de de Jean-Marc Boyer, que nous avons déposé effectivement dans la suite de la mission d'information, je l'ai dit tout à l'heure lors de mon avis sur le budget, c'est la deuxième année, première années où vous aviez annulé les 110 ETP qui devait disparaître et la deuxième année où vous effectivement vous stopper l'hémorragie, vous créez 15 ETP sur le médico-social mais nous souhaitions avoir quand même cette alerte et cet amendement pour vous dire que nous serons très vigilants parce que l'enseignement agricole demande une pédagogie par petits et donc cela va nécessiter de pouvoir recruter des enseignants supplémentaires mais vous nous avez vous êtes engagé lors de l'audition que nous avons mener effectivement sous la présidence de Laurent Lafon à nous tenir au courant de plan pluriannuel que vous allez négocier sur les ETP, donc voilà, je retire donc cet amendement parce que vous vous êtes engagé effectivement à nous tenir au courant et que vous avez je pense compris l'alerte. Le quatre cent cinquante est retiré Monsieur Besson. De de mots sur sur l'ensemble de ces amendements, d'abord vous remercier monsieur le Ministre de votre présence, c'est la première fois, lors du débat de la mission scolaire que nous avons le ministre de l'Agriculture, votre prédécesseur monsieur éducation nationale a eu des moments beaucoup plus difficile, nous ne pouvons pas toujours répondre à nos questions et votre présence est une marque importante pour le Sénat de deuxièmement je voudrais dire qu'il y a Monsieur le Ministre, Éducation nationale, certainement, à regarder ce qui se fait alors dans l'enseignement agricole en matière d'enseignements généraux dans la voie professionnelle au moment, vous envisagez de réformer la voie professionnelle, il y a certainement beaucoup à apprendre en matière de place d'enseignement général dans cet enseignement largement professionnel et en particulier comme vous l'avez dit, monsieur le Ministre, la qualité de l'enseignement dit socio-culturels qui est certainement n'a enseignement civique de grande qualité, même s'il n'importe pas le nom parce que les propos, monsieur, puis il a dit, on ne parlait pas tout à fait aussi. Merci madame Billon. Merci monsieur le président, donc moi je, je me félicite des annonces et et des réponses qui ont été données par le le ministre de l'Agriculture et sa présence évidemment ce soir, je me suis permis Monsieur le Ministre, comme j'avais 8 minutes dans la discussion générale, de vous faire part de cette, de ce cas particulier, tout à l'heure parce qu'il dénotait quand même un problème important dans la manière de, de, de gérer les ressources humaines d'une ministère vous y avait répondu ce soir et je vous en remercie, je vais pour ma part, retirer les, les, les amendements puisque j'ai les réponses à mes questions, la seule chose, c'est que je disais que il n'y avait pas d'horaire dédié dans certaines classes de l'enseignement agricole pour ces matières là et donc voilà, c'est une réponse qui peut être peut être pourra être creusé un peu plus, merci pour votre présence et merci pour ces réponses et je retire mes amendements oui merci Monsieur le Président, eu égard à ce qui a été dit à la fois par le rapporteur, et bien sûr les réponses apportées par le ministre, je retire mes deux amendements. Très bien, donc le sont retirés à ce stade de 234 le 450 le 600 hein le 235 et le six je vais faire voter sur les autres amendements des 2 amendements identiques: le 800 76 et 941 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté même vote pour le 941 même vote il n'est pas adopté même vote pour 942

pas adopté le 939 même vote pas adopté de 882 même vote pas adopté. Alors, mes chers collègues, il est quasiment minuit il nous nous reste 3 quarts d'heure pour faire vingt-cinq amendements. Donc, et on doit tenir les délais, donc il y a rien d'impossible, mais il faut faire court, y compris Monsieur le Ministre. Voilà donc, nous passons 454 la présidente de. Oui, merci, c'est un amendement qui est co-signé par une cinquantaine de sénateurs et qui fait suite, notre mission d'information avec le le président Boyer, mission d'information, qui avait fait de nombreux constats notamment l'excellence de l'enseignement agricole, sa qualité pédagogique ses taux de réussite, son taux d'intérêt Serge Sion bien plus haut que que la moyenne générale et des filières générales, mais des métiers que les Français, donc les jeunes ne connaissent pas, avec donc une préconisation forte sur la communication, qui permettrait une reconnaissance, mais surtout une connaissance de de de ces filières et de ses métiers, alors qu'on sait qu'il y a urgence à intégrer ces filières pour notre souveraineté et notre résilience alimentaire, je l'ai dit tout à l'heure dans la discussion générale 10 millions avaient été mises avait été mis pour lancer la communication, il y a 2 ans avec le camion du vivant, le camion orange avec beaucoup de communication, c'est un point de divergence qu'on avait un pont dans le l'audition, nous avions quand même un sentiment général de ne pas avoir véritablement vu de commission communication cette année vous en étonnez un peu mais c'est un sentiment c'est un ressenti quand même très fort, c'est pour ça que nous sommes plusieurs à vous présenter cet amendement pour augmenter les Budgets de la communication pour rendre visible cet enseignement qui nous est indispensable. Chers collègues, mais si on fait une minute 30 par présentation, je vous assure qu'on ne tient pas la route, hein, on ne tient pas la route. Ah oui, monsieur le Ministre. Pardon, monsieur le rapporteur de Laborde excusez-moi hé bien le rapporteur est favorable, il n'y a pas d'amour sans. Preuve d'amour et ça vraiment s'en prend pour de briques, mais ça permet d'apprendre, d'affirmer notre soutien d'enseignement agricole et à sa promotion si Monsieur le Ministre. monsieur le président, c'est une demande de retrait sinon défavorable, parce qu'au fond, madame la présidente, vous disiez et Madame la rapporteure, néanmoins, vous disiez : on en a parlé en commission, c'est un objet de désaccord, il me semble que on peut pas à la fois dire on ne sait pas trop ce que j'ai fait des moyens parce que vous parlez des des du budget 2022 dire il faut rajouter des moyens, il me semble qu'il y a quelque chose qui est un peu contre-intuitif, en tout cas pour moi et donc c'est une demande de retrait sinon des défavorable mais en revanche, je vous l'ai dit en commission, on va faire une analyse précise de ce qui a été l'utilité mais au fond il y a que le résultat qui compte, ce que je constate cette année c'est qu'il y a plus d'élèves dans l'enseignement agricole et que peut-être, même si vous ne l'avez pas vu il y a des gens qui l'ont vu, par ailleurs, je signale qu'avec mon collègue PAP Ndaye on a fermement l'intention de travailler sur les questions d'orientation de présentation des métiers agricoles, il pourrait dire mieux que moi, mais comme j'ai le micro pour l'instant et ruraux et ruraux rapporteur raison de le dire, merci.

Merci monsieur le président, donc c'est un amendement qui fait suite au rapport rédigé par nos collègues Cabanel et Françoise Férat sur les suicides en agriculture, c'est un amendement qui propose d'intégrer au programme des modules relatifs à la à la connaissance, indicateurs de bien-être, une prévention du burn-out mais aussi une formation aux tâches administratives que les jeunes ne quantifie pas comptabilité évaluation des normes environnementales procédure demande d'aide propose donc en conséquence d'augmenter les crédits d'enseignement technique agricole un millions d'euros. Merci, monsieur le rapporteur. Défavorable, c'est une formation qui est déjà délivrés par les établissements ce ministre. Pour les mêmes raisons, c'est le d'un avis défavorable, simplement je reconnais le travail volontiers, qui a été fait par le sénateur Cabanel, sa collègue et le c'est le député de la maison qui travaille beaucoup sur ces questions de mallettes alors c'est il y a des choses qui sont délivrés dans les dans ce lycée d'enseignement, je ne peux pas m'arrêter quelques instants sur la situation de mal-être, il faut dire qu'il y a une mission qui a été confiée, il y a quelques temps dans le cas de du plan de lutte contre le suicide et le mal-être dans l'agriculture, qui sera prolongée, je vous le, je peux vous le dire ce soir dans les mois qui viennent, à l'issue de celui qui est missionné actuellement parce qu'on a besoin de travailler sur ces sujets-là et d'accompagner que on ait une vigilance particulière, département par département, sur ces questions de ma lettre, mais pour ce qui est l'enseignement agricole, les choses sont faites me semble biotine sérieusement. Si jamais il est retiré, il est retiré de 776 2 amendements en discussion commune le 886 madame. Oui, monsieur le président, malgré des efforts depuis plusieurs années pour amener le coût de la rémunération des assistants d'éducation, de l'enseignement agricole au niveau de celui de l'éducation nationale le PLF 2023 continue à amplifier l'écart à 580 euros par agence, soit 728070 euros écart cumulé à remettre à niveau à niveau au regard du PLF 2023, de l'éducation nationale, à noter que le salaire des agents étant le même qu'il soit l'éducation nationale ou en lycée agricole du fait de la différence de crédit, ce sont les établissements agricoles qui sont contraints de rémunérer sur leurs fonds propres ou parfois de limiter l'emploi d'assistants d'éducation, compromettant l'encadrement et la sécurité des élèves à cet amendement vise donc à porter les crédits au titre des personnels assistants d'éducation, de l'enseignement agricole agneau hauteur équivalente de ceux du ministère de l'Éducation nationale. merci, monsieur le rapporteur, la commission a demandé le retrait, moi je demande l'avis du ministre merci monsieur le Ministre. Oui, monsieur le président, monsieur le rapporteur, c'est une demande de retrait, sinon c'est un avis défavorable, effectivement, il y avait un écart qui avait été faits, je vous rappelle que vous aurez noté que, il y a un effort qui consiste à bander de 3 virgule 36 millions d'euros les crédits dédiés à la rémunération, l'idée c'est de converger, on est quasiment à l'alignement, et donc il me semble que on est en train de satisfaire ce que vous avait demandé donc c'est une demande de retrait six non, c'est un avis défavorable. Merci sont maintenus. je mais aux voix le 886 avec 2 avis défavorables. Qui est pour, qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté même vote pour 943, il n'est pas adopté le 1256 du gouvernement Monsieur le Ministre. monsieur le président, Mesdames et messieurs, le rapporteur je train de le faire à deux voies avec mon collègue ministre de l'Éducation puisque c'est sur les après les échanges que nous avons eu que nous vous faisons ces propositions d'amendement qui vise à abonder de 566000 5000 euros la ligne budgétaire dédiée au programme enseignement technique agricole pour augmenter de 50 les crédits dédiés au fonds social lycéen ça avait été dit d'ailleurs par votre rapporteur sur ce sujet, l'objectif est, et qu'on on essaye de d'intégrer le dispositif dans le cadre de l'enseignement agricole et donc voilà l'amendement qui vous est proposé, ça permettra d'apporter un soutien accru aux familles en difficulté, quel que soit le mode d'enseignement, y compris l'enseignement agricole. Si monsieur le rapporteur. Commission n'a pas eu le temps de d'examiner cet amendement, qui est arrivé tardivement spontanément, j'émets un avis favorable en rappelant cependant Monsieur le Ministre, ce que souvent les fonds sociaux ne sont pas utilisées.

sous encore une fois la la houlette du président font on nous avions alerté sur cette problématique et ce petit dysfonctionnement et donc nous sommes ravis que vous répondiez aussi vite par un amendement pendant la la discussion merci, ministre de l'éducation, de permettre de rétablir ce compte.

Merci, Monsieur le Ministre, n'a pas la réponse. 230. Voilà donc je mais voit cet amendement du gouvernement le 1256 à favorable du rapporteur. Qui est pour, qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté 2 amendements en discussion commune 940 madame brûlant. Merci monsieur le Président, c'est un amendement qui propose de revaloriser l'ensemble de la grille indiciaire des AESH au sein de l'enseignement technique agricole je ne reviens pas sur les inégalités qui ont été développés avec leurs collègues de l'éducation nationale, je ne reviens pas non plus sur le chiffre qu'a donné la rapporteure Nathalie Delattre tout à l'heure sur une augmentation de 26 % des élèves en situation de handicap dans l'enseignement agricole qui montre les besoins d'accompagnement qu'il y a et si au 1er mai 2022 les deux premiers échelons de la grille indiciaire des oeufs va E H ont été revalorisé pour atteindre le niveau du SMIC, ça n'a pas été le cas pour les autres échelons, ce qui entraîne un tassement de la grille préjudiciable à nos yeux. 884 de ce entraîne. Oui, merci Monsieur le Président, je souhaite, chers collègues, attirer votre attention, justement sur la situation particulière des AESH exerçant dans l'enseignement agricole et maritime au nombre de 700 environ, ils sont confrontés à des conditions d'emploi encore plus difficile, quantité de travail comprise entre 10 % et 20 % non accès aux dispositifs de formation, si bien qu'ils se qualifient eux-mêmes de sous à ESH alors par équité vis-à-vis de l'ensemble des personnels Osh, cet amendement vise la revalorisation des des échelons de plus de 15 points minimum sur l'indice brut afin que ça hausse soit répercutée le coût estimé est de 32737 euros pour cette valorisation. Monsieur le rapporteur. Défavorable dans les 2 cas et nous renvoyant la réflexion globale sur les avis sèche. Merci, monsieur le Ministre.

il me il me semble qu'il faut faire attention parce que je trouve que le travail qu'ils font remarquer a, par ailleurs, on a, on l'a dit avec mon collègue ministre de l'éducation, il l'a dit avant moi, on est en train de faire converger les grilles, donc on est sur les mêmes dispositifs par ailleurs vous dire que dans la période 2017, 2022 on aura quasiment tripler le nombre d'AESH et on répond aussi à la demande, ça a été dit par le sénateur Brisson, d'ailleurs, il y avait beaucoup de retard, tout le monde doit prendre sa responsabilité, il y avait beaucoup de retard d'accumuler, on essaye de prendre la part de rattrapage de retard sur ce sujet donc demande de retrait sinon défavorable. Merci donc je mais aux voix ces deux amendements tout d'abord le 940 avec 2 avis défavorables. Qui est pour, qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté de 884 même botte mais vote il n'est pas adopté de 913 du président le jour. Oui, merci Monsieur le Président, cet amendement vise à inciter à l'organisation de sorties scolaires régulière de découverte de la nature de l'école, au lycée, cela pourrait prendre la forme d'une demi-journée scolaire en extérieur sous forme de sortie éducative hebdomadaires ou bi-bimensuels, afin de sensibiliser les jeunes générations à la préservation de la biodiversité et à la découverte de la nature conserver au recréer du lien entre les jeunes et les espaces naturels proches est un des enjeux majeurs pour réussir la transition écologique dans les prochaines années, et si l'on veut permettre aux plus jeunes, de mieux comprendre comment protéger l'environnement, il est à, il est essentiel et indispensable d'intégrer la reconnexion au vivant comme élément clé dans les programmes scolaires, c'est pourquoi nous proposons que chaque établissement scolaire de l'école primaire au lycée, développe un projet de sensibilisation à la biodiversité et une telle mesure doit permettre de sensibiliser les élèves à ces gens, à l'échelle locale en les impliquant directement en tant qu'acteur pour agir pour la bio diversité, je vous remercie. je ne suis pas certain qu'elle soit complètement mûri dans son dispositif, et puis alors que faire pour les jeunes ruraux, on pourrait aussi les emmener en ville parce qu'ils ne connaissent pas le monde urbain et je pense qu'il faudrait évoquer cela également. Merci, monsieur le Ministre. Même avis que le rapporteur spécial avis défavorable. Merci Monsieur président bonjour. Ben, je vais le retirer mais c'est un amendement d'appel quand même parce qu'il faut, on peut pas parler de, de, d'environnement, tous les jours, on peut pas parler de biodiversité, le matin, le midi et le soir et puis que on sensibilise pas les plus jeunes d'entre nous je le redis. Merci de ne 48 Merci monsieur le président, tellement je m'excuse auprès des 33 cosignataires qui ne figure pas sur le document il y a eu un problème de communication avec la séance dont j'assume la responsabilité, amendement, il concerne et 70 pour 100 d'élèves qui relève de l'éducation prioritaire, scolairement et socialement, mais qui ne bénéficient pas de ces moyens, tout simplement parce qu'ils sont sur des territoires oubliés

lorsqu'elle fait fonctionner l'ascenseur social pour le faire fonctionner, on a créé dans les années 90 des heures zone puis après des réseaux d'éducation prioritaire 2014, 2015, il y a une réforme qui va complètement bouleverser le système en a incluant un critère d'éligibilité géographique avec le lien avec un quartier politique de la ville qui va complètement exclure les zones rurales et de nombreuses zones urbaines, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a trop de gamins qui relève de s'éducation prioritaire qui n'y sont pas le ministère votre prédécesseur et vous-même êtes conscient de cette problématique et des experts expérimentation pardon ont été créés les territoires éducatif ruraux et les contrats locaux d'accompagnement très bien, sauf qu'ils sont dotés, très peu 9 millions d'euros, il faut une vraie réforme, elle est annoncée, elle est attendue, elle est différée depuis des années, alors avant de faire la réforme de façon palliative, je vous propose de d'abonder de 10 millions d'euros crédits doté enfin ces crédits pour ces territoires qui en ont besoin lors de ce que vous êtes venus devant la commission Culture vous êtes vous avez vous-même reconnu qu'il fallait effectivement réformer cette carte et donner plus de moyens à tous ces territoires, c'est ce que je vous propose par cet amendement. Hé, chers collègues de la concision, monsieur le rapporteur. Oui, j'ai le président là, la commission des finances, est très intéressé par ce travail, cette réflexion conduite par notre collègue Olivier Paccaud mais c'est une affaire très récente, puisque l'extension date de septembre 2022 étendue à cette nouvelle académies, vous l'avez si signalé et c'est peut être un petit peu tôt pour prendre une décision aussi forte que cet abondement de 10 millions d'euros, donc notre idée plutôt le retrait, on devrait avoir le sentiment du ministre. Monsieur le Ministre. Monsieur le président, monsieur le rapporteur spécial, en effet, nous sommes encore dans une phase d'expérimentation puisque les classes sont déployés dans 5 académies les territoires éducatif ruraux dans 10 académies, il y en a actuellement 67, il nous semble donc l'enveloppe actuelle et et calibrée aux besoins de l'année 2023, à ce titre-là d'expérimentation j'émets donc un avis défavorable à votre amendement. Merci donc je ne sais pas quo. Non je je ne le retire pas mais je suis quand même déçue parce que il n'y a plus de secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, il en a plus dans votre gouvernement et là cette c'est le seul moyen de de rééquilibrer un petit peu cette problématique alors 10 millions d'euros, ça paraît beaucoup, mais des millions d'euros sur 59 milliards le budget de l'Éducation nationale, excusez-moi, c'est une paille alors que c'est, c'est un symbole très fort donné en faire ces territoires qui sont oubliées,

Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté 4 amendements identiques le 63 madame Darcos. Merci monsieur président cet amendement de notre collègue Philippe mouiller vise à octroyer les moyens supplémentaires à l'éducation nationale pour permettre à chaque enfant en situation de handicap d'avoir accès au matériel pédagogique adapté, reconnu comme nécessaire à son par car à son parcours de scolarisation par la par la CDA à Ph de nombreux parents font état, difficultés pour que leurs enfants puissent bénéficier de ce matériel pédagogiques adaptés pourtant notifié par la CEDEAO PH, il aurait souvent répondu que par les services académiques que les crédits annuels seront épuisées et qu'il leur faudra attendre l'année prochaine, dans un contexte où le gouvernement entend faire de l'école inclusive une priorité cette réalité n'est pas acceptable et mais de nombreux élèves en difficulté car en défaut d'autonomie. Oui, tout à fait de la politique pour l'école inclusive, c'est des moyens en matière d'AESH c'était évident de statut des AESH mais aussi en matière de matériel, notamment informatique destiné aux élèves qui en ont besoin et il y a une carence très forte, plus de 21000 gamins qui n'en ont pas actuellement et qui en auraient besoin. Merci de 453. Défendu le 874 défendu aussi, monsieur le rapporteur. Sur ces quatre amendements identiques

Merci, monsieur le Ministre. au budget précédent à quoi s'ajoute le fonds d'innovation pédagogique puisque des projets pédagogiques pourront en effet servir à l'achat de ce matériel, compte tenu de ces éléments, j'ai émis un avis défavorable à ces propositions, dont bien entendu je partage la philosophie générale. Merci donc je vais mettre aux voix les quatre amendements identiques 63 203 453 874 avec 2 avis défavorables. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés. 2 amendements en discussion commune de 275 et 276 Monsieur Bresson. Bresson. Le président je vous propose de présenter les deux très rapidement, 2 amendements d'appel mais qui pose de vrais problèmes de constat 1er constat notre école n'assure plus la transmission des savoirs fondamentaux, les classements internationaux l'la dégradation et continue 2ème constat notre école n'assure plus l'égalité des chances, c'est une école de la non-mobilité sociale, c'est même un record en Europe pour réagir, une proposition d'amendement 200 francs de quinze propose de créer un service public de soutien scolaire et l'amendement 276 une réserve éducative pour mettre en oeuvre ce service public. Merci, monsieur le rapporteur. Là aussi je suis écartelé entre l'avis de la commission que je rapporte avec fidélité, qui est une demande de retrait et puis le fait que je suis co-signataire de cet amendement, ce que vous pouvez d'ailleurs constaté juste après Max Brisson, qui m'a donné cette excellente idée, ne serai pas plus long, on va prendre l'avis de la commission donc retrait ou défavorables. Monsieur le Ministre. Oui le le dispositif d'aide au devoir est abondé au PLF 2023 à hauteur de 81 millions d'euros, je rappelle que plus de 800000 élèves ont bénéficié de ce dispositif, soit 30 % de l'ensemble des collégiens, ce qui nous semble être significatif et également correspondre ou demandes exprimées par les collèges et donc pour ces raisons, j'émets un avis défavorable. Merci Monsieur Bresson. Monsieur le président, pour ne pas mettre notre rapporteur spécial dans l'embarras : je vais retirer ces amendements mais on est au fond du sujet : le problème il est majeur : la dégradation de la transmission des savoirs fondamentaux s'accélère donc de Vienne humiliant. Notre situation donc est extrêmement inquiétante et en matière de mobilité sociale nous sommes cancre, seules la Hongrie fait plus mal. Donc, aujourd'hui, il faut réagir et une politique de moyens supplémentaires et de rustines en termes de réorganisation profonde du système ne fonctionne pas, donc nous avons posé ces amendements, nous y reviendrons, je pense que vous ne sortirez pas de cette situation extrêmement dramatique pour le pays sans de véritables réformes de fond, les de propositions qui étaient sur la table sont des réformes de fond. Merci donc ils sont retirés le 598 madame Mabillon. donc je vous avez le l'objet sous les yeux, je vous laisse lire et et on va gagner du temps, puisque c'était demandé par le président. Si, si, monsieur le rapporteur et du Gouvernement avait du gouvernement Monsieur le Ministre.

de celle où se situe son institut de formation ou bien il y a la possibilité d'indemnités kilométriques qui bénéficie aux stagiaires et par ailleurs, les contractuels, alternant, dans le cadre des formations Metz de de master perçoivent depuis le 1er septembre 2022, une indemnité de 700 euros brut annuels pour compenser leurs frais de déplacement entre leur lieu de des, de formation et l'établissement où ils exercent compte tenu de ces éléments et de ces évolutions mises en oeuvre, je suis défavorable à votre amendement. En fait, je vais le maintenir parce que c'est vrai que, il y a des efforts de faits, mais cela ne semble pas suffisant pour rendent toujours attractif et on le voit, il y a des démissions, donc je le maintiens. Pour la forme, donc je le mets aux voix avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 891 monsieur entraîne. Oui, Monsieur le Président, cet amendement, il vise à augmenter le nombre de classes Ulis dans les écoles du second degré, par exemple en 2021, on a presque un enfant sur 5 qui n'a pas pu être scolarisés dans l'environnement, faute de places suffisantes ainsi le nombre de prescriptions de scolarisation en classe Ulis augmente, il est nécessaire d'augmenter la la, à la même vitesse, les places en classe Ulis ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le taux de couverture des notifications est en baisse, ainsi, cet amendement vise à réduire ces situations d'impasse qui parfois oblige les familles à sortir leurs enfants du système scolaire public pour se diriger vers une instruction en famille, faute de possibilités d'accueil adapté. La commission demande l'avis du gouvernement, parce que nous n'avons pas eu le temps dans le délai imparti de l'approfondir la question. monsieur le président, nous avons plus de dix 10000 dispositif Ulysse, il est prévu la création de 300 dispositif Ulysse au PLF 2023, ce qui représente un effort de 336 ETP supplémentaires, c'est donc tout à fait conséquents je rappelle, par ailleurs, la réflexion que nous de fond que nous menons dans le cadre de la préparation de la conférence nationale du handicap qui se prépare pour le printemps 2023 pour ces raisons, j'émets un avis défavorable. Merci donc je vais au bois 891 avec 2 avis défavorables. C'est pour qui est contre. Il s'abstient, il n'est pas adopté de 917 Madame de Marco. Oui, l'éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire des enfants est inscrite dans la, dans un article du code de l'éducation, c'est donc une obligation, mais celles-ci ne bénéficient pas d'heures d'enseignements dédié ce présent amendement vise à créer un fonds pour permettre aux établissements de mettre en place des projets d'éducation à l'alimentation. Merci, monsieur le rapporteur. Commission en à deux demande le retrait de cet amendement parce que d'une part, beaucoup d'efforts sont déjà faits par les enseignants eux-mêmes, d'autre part 2 millions ne changeront pas la face du monde, compte tenu du nombre d'élèves concernés. Ce ministre-même avis. Même avis monsieur le le président j'ajoute à cette l'argument du rapporteur spécial, le fait que les crédits pédagogiques qui sont mis à disposition de tous les établissements permettent de tels enseignement auquel je suis évidemment favorable donc avis défavorable sur l'amendement.

l'agroforesterie est une tactique qui associe les arbres à la production agricole, cultures et élevage au sein de parcelles agricoles cette technique qui est ancestrale se pratique par la plantation de haies autour de parcelles ou de manière inter-parcellaire, c'est-à-dire par la plantation d'arbres en alignement, l'objectif est à la fois économique et écologique en effet l'agroforesterie permet d'améliorer les rendements agricoles de manière significative, elle lutte contre l'érosion des sols, elle permet la production de bois et donc de diversifier les revenus de l'exploitation, les arbres Servent également d'abri pour les animaux, limite le ruissellement et contribue à la préservation des paysages, le développement de l'agro-foresterie sur les territoires français ne peut se réaliser que par la formation des agricultrices et des agriculteurs ainsi que grâce à l'aide des conseillers techniques afin d'augmenter le nombre des conseillers et conseillères agro- forestier au sein des chambres d'agriculture, la création d'une nouvelle formation en agroforesterie est nécessaire, alors qu'il existe des formations gestion forestière la formation spécifique à l'agroforesterie existantes, cet amendement propose donc la création de 15 nouvelles formations BTSA en agro-foresterie. Merci monsieur le président, monsieur le rapporteur spécial mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le, c'est le président, simplement pour vous dire quand vous regardez le, les métiers de l'agroforesterie ça vient souvent des métiers de des forestiers, hein, c'est de là qu'est partie l'agroforesterie, vous avez raison et vous avez souligné qu'ils étaient d'intérêt de l'agroforesterie, ce que je peux vous dire c'est que déjà que l'enchaînement de synthèse, cette technique est intégré dans la au cursus BTSA Gestion forestière dans lequel il y a l'agroforesterie et les autres métiers de la forêt vous a indiqué en août que nous avons ouvert 2 sections supplémentaires, ce qui fera qu'on ça viendra s'ajouter au 34 BTSA qui permettent de traiter de ces questions forestières et donc d'agroforesterie et donc le mon nombre de places vacantes diminue chaque année mais le dispositif actuel suffit accueillir davantage de d'étudiants, et donc je vous demande un retrait, sinon c'est un avis défavorable, les choses étaient ont déjà posé l'agroforesterie étant évidemment déjà enseigné dans un paquet plus globale autour du forestier. Merci, monsieur le Ministre, monsieur. Monsieur le Président, compte-tenu des explications du midi je retire cet amendement. 912 et retiré de 919 Madame Meunier. Merci donc je parle au nom de Lucien sur cet amendement vise à prévoir la mise en place d'une expérimentation dans l'académie d'Aix-Marseille d'orthophonie accessible à l'école pour les enfants des classes Ulis des écoles du 1er degré hors intervention déjà réalisé dans le cadre des services d'éducation spécialisée et de soins à domicile aujourd'hui les enfants des classes Ulis des territoires ruraux doivent prendre un taxi et père d'une matinée d'enseignement pour se rendre chez l'orthophoniste, alors qu'ils sont déjà en grande difficulté au niveau des apprentissages, les inégalités territoriales perdure, voire s'accentue avec les effets de la crise Covid auxquels se rajoutent les conséquences de la crise ukrainienne construire l'école inclusive de demain, nécessite de renforcer le travail partenarial entre les professionnels de santé sociaux et d'éducation, il en va de l'égalité des chances pour les élèves des classes Ulis qui nécessitent des besoins spécifiques pour une meilleure progression intégration dans leur vie active futur scènes une société plus plus plus inclusive, développer des prises en charge au sein de l'école serait par ailleurs une bonne solution pour réduire la fatigue des élèves et prendre en plus enfin en charge, notamment dans les milieux défavorisés. La Commission estime que cette n'est pas d'ordre législative donc refus retrait pardon. Monsieur le Ministre. C'est le président de la les orthophonistes, madame la sénatrice Monnier les orthophonistes peuvent d'ores et déjà intervenir au sein d'un établissement scolaire, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expérimentation j'aimais donc un avis défavorable à cet amendement.

Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, il y a quelques semaines, j'ai reçu un groupe de parents, d'enseignants, de CPE d'élèves totalement abasourdi et indigné par la décision qui venait de découvrir, en pleines vacances de la Toussaint, de la fermeture pure et simple à la rentrée prochaine de cet établissement à Paris 6, lycée professionnel et un lycée général qui met en oeuvre des formations artistiques dans le spectacle vivant et la danse assez unique, cette décision va en plus impacté les 20 établissements qu'on oblige à accueillir les élèves qui perdent leur établissement à la rentrée prochaine, c'est une décision incompréhensible mais le pire c'est que la justification, ce qui explique la forme de l'amendement, la justification de cette décision, c'est de faire une économie de sobriété énergétique, donc c'est la facture énergétique de ces établissements qui justifierait leur fermeture, ce qui est quand même assez incroyable quand on parle de sobriété énergétique, il y en a qui traduisent à la région Île-de-France, fermeture de lycée professionnel, alors j'aimerais savoir Monsieur le Ministre, pourquoi le ministère a laissé faire et soutien de fait, cette décision, d'autant que, visiblement, la région Île-de-France, laisse entendre qu'elle procédera chaque rentrée prochaine à une vague de fermetures de lycée professionnel à Paris. Monsieur le rapporteur. Demande de retrait parce que n'étant pas de compétences. Monsieur Ministre. Monsieur le président, monsieur le sénateur, les le les 2 explications sont les suivantes : le contexte de baisse démographique accéléré à Paris, deuxièmement la vétusté des locaux, nous nous assurons du côté du rectorat, de même que du côté du ministère de l'éducation nationale, que ces transferts et ces fermetures ne provoque aucune dégradation de l'offre de formation, je m'en suis assuré moi même, je peux même vous dire qu'il y aurait une amélioration en réalité de l'offre de formation quant aux fermetures et au transfert il s'effectue dans des secteurs géographiques qui n'impacte pas la scolarité des élèves concernés, tout au contraire : avis défavorable. mais Monsieur le Ministre, on passe d'établissements à taille humaine de petits établissements qui accueillent accueille un public populaire et vous les mettez dans les établissements de 2000 élèves et vous dites que ça change rien alors qu'en plus ce sont des formations spécifiques, alors moi je vous conseille de recevoir les parents et les enseignants qui vous demande depuis plusieurs semaines, d'être reçus pour vous expliquer la situation de ces établissements. je mets au bois de 931 avec 2 avis défavorables. Qui est pour, qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 889 ma Monnier. Donc, cet amendement vise à abonder de 390000 euros les crédits en faveur des subventions aux associations assurant la mise en oeuvre des politiques éducatives, plus particulièrement en charge l'accompagnement de l'éducation à la vie affective et sexuelle, ces subventions ne doivent être. Revalorisé a minima au niveau de l'inflation, l'éducation à la vie affective et sexuelle est un apprentissage fondamental qui doit être inclus dans le cursus scolaire à tous les niveaux, c'est ce que Didier était décidé dans la loi Aubry de 2001 qui a été réaffirmée en 2018 par la circulaire Schiappa à raison de 3 séances d'éducation à la sexualité par an et par niveau dès le plus jeune âge, malgré l'inscription dans la loi, on constate que l'éducation est très parcellaires, quand elle n'est pas totalement inexistante dans certains établissements et les établissements scolaires sont demandeurs, chaque année, des mais les de d'association comme le planning familial, mais ils sont contraints de refuser parce qu'ils n'ont pas assez de moyens il a vraiment urgent, a changé la donne, je rajouterai que, dans les milieux défavorisés l'information délivrée par les structures publiques associatives sur ce sujet est souvent la seule que reçoivent les élèves issus de ces territoires, hormis celle totalement déformée inadaptés que leur transmettre les réseaux sociaux, l'éducation à la sexualité constitue aussi un enjeu de santé publique information. Sur la grossesse non désirée, sur les maladies sexuellement transmissibles ou les conséquences dramatiques sur la santé mentale des violences sexuelles et sexistes. Commission un avis défavorable, considère que n'est pas l'éducation nationale, de financer des associations dont personne ne connaît l'orientation ou le genre.

et d'autre part que c'est aussi à l'école, elles-mêmes, d'assurer l'éducation à la sexualité, par ailleurs, ces associations ne couvre pas l'ensemble du territoire, donc nous avons à ce à nous saisir nous-mêmes de cette obligation légale et de cette obligation, pour les raisons que vous avez indiqué, j'aimais donc un avis défavorable à cet amendement, tout en partageant bien entendu l'objectif que vous indiquez. Si Madame Monier. Juste, Monsieur le Ministre, les associations quand elles sont sur le terrain qu'elles peuvent le faire, il faut leur donner des moyens supplémentaires, je pense que c'est essentiel et j'ai du coup j'ai perdu la 2ème idée je prie parce que. Y'chers collègues je mais on voit le 800 89 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, je demande à chacun de se préparer, parce qu'il va y avoir un scrutin public qui a été demandée par la Commission sur les crédits de la mission alors, nous passons à l'amendement 673 Madame de Marco. Même si cet amendement d'appel à pour l'objet la création de nouvelles enseignement des enjeux de la protection sociale et environnementale, le rapport d'information construire la sécurité sociale du XXIe siècle porté par notre collègue Mélanie Vogel recommandé d'ailleurs une meilleure formation sur les Liens entre santé environnement en fin de passer d'une logique de traitement, une logique de prévention, il importe que le plus tôt possible, les jeunes qui seront les adultes de demain comprennent la gravité du changement climatique, il les aime pas corrompre sur leur santé, si risque afin de leur donner les clés de réflexion une mobilisation personnelle sur ces enjeux.

alors le rapporteur pourrait se réjouir. Que voilà un amendement à un euro. Bon, à tout prendre, si ça peut vraiment faire plaisir mais honnêtement, je pense que l'éducation nationale est parfaitement tant en mesure d'assurer la culture et l'ouverture de nos jeunes élèves sur les réalités, dans la mesure des programmes qui sont les siens de l'économie de l'histoire de l'histoire sociale, d'une certaine façon, enseigner les enjeux de protection sociale et environnementale pour un Euro, je ne vois pas très bien ce à quoi ça correspond et c'est la raison pour laquelle je suggère le retrait, j'en profite pour dire parce que vous avez évoqué le le scrutin qui va intervenir après ce dernier amendement, on est bien d'accord, à ma connaissance, mais je ne suis pas ma compétence n'pas universellement peut parfois être étonné la commission n'a pas demandé ce que as un public pardon Union centriste, je me suis trompé le groupe Union centriste. Il a demandé voilà tout à fait, je me suis trompé, excusez-moi, monsieur le rapporteur. Alors je, je, je, j'indique simplement à nos collègues qu'on peut adopter ou rejeter le budget. Mais si on le rejette tous les amendements que nous avons examiné son disparaissent, donc nous aurons en quelque sorte en termes vulgaires pisser dans un violon pendant 3 heures. Monsieur le ministre, alors nous restons sur l'amendement 673 nous restons son amendement 673, monsieur le ministre. Monsieur le président, Monsieur le rapport spécial même même avis que monsieur le rapporteur spécial quant à son analyse de l'amendement concernés : avis défavorable. Madame de Marco. C'était un amendement d'appel je le retire. Qu'il ait retiré 673, sur les, les, les crédits de la mission et j'étais donc du saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Union centriste avec un avis de la commission qui est favorable, il va être pour procéder au scrutin public le scrutin tout ouvert.

La demande à voter. Plus personne, le scrutin est clos.

Nous passons article additionnel après l'article 43 le 223 monsieur Grosperrin.

vers le premier degré, car à ce jour dans le 1er degré, il y a pas de Canal, justement, qui permet de versements aux établissements des crédits qui accompagnent un certain nombre de politiques dont les crédits d'innovation pédagogique la les territoires éducatif ruraux, ces derniers n'étant pas autorisés à recevoir des crédits pédagogiques, donc c'est simplement un canal qui va simplifier les choses et qui permettra aux établissements du 1er degré de pouvoir avoir ces produits-là. favorable, Monsieur le Ministre. et en 1er Lyon au fonds d'innovation pédagogique, je suis donc favorable à votre amendement. qui est contre. Qui s'abstient, il s'il est adopté et enfin d'amendement 1181 de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, c'est un amendement qui a pour objet après l'article 43 d'insérer un article additionnel, les conditions d'attribution de la prime de rémunération, c'est-à-dire le pacte accordée aux enseignants, au titre de la réalisation de missions supplémentaires sont définies par décret avant le 31 mars 2023 c'est un amendement d'appel pour dire simplement qu'on aimerait bien que l'argent du pacte soit que équilibré et connu de la représentation nationale et du Parlement avant les cas dans Mirek si Monsieur le Ministre. Monsieur le président, monsieur le rapporteur spécial, tout en partageant ce que vient de dire le rapporteur spécial, je me suis engagé à ce que cette revalorisation intervienne en septembre 2023, c'est cet objectif qui guident notre calendrier et je peux vous dire que cet objectif sera tenu dès lors j'émets un avis de retrait de cet amendement, sinon, sinon un avis défavorable. et on aimerait connaître les contreparties donc je le retire, mais avec une une question d'actualité qui sera posée à cette date. Merci, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance vendredi 2 décembre à 9 heures 45 pour l'examen de la mission cohésion des territoires du projet de loi de finances pour 2023 à la séance est levée.